monsieur le président

La séance est ouverte. Le compte rendu intégral de la séance du mercredi 31 octobre

Je rappelle au Sénat que le groupe socialiste et républicain a présenté la candidature de Mme Hélène Conway-Mouret pour remplacer, en qualité de vice-présidente du Sénat, Mme Marie-Noëlle Lienemann.

je proclame Mme Hélène Conway-Mouret vice-présidente du Sénat, et je lui souhaite pleine réussite dans l'exercice de cette fonction éminente au sein de notre assemblée. Je tiens à remercier Mme Marie-Noëlle Lienemann pour sa vice-présidence. Elle a présidé nos travaux avec une qualité d'écoute reconnue par chacun et une maîtrise parfaite de nos règles de procédure. J'ajouterai un sentiment personnel,

qui veillent à l'expression de tous les sénateurs et à la qualité de nos délibérations et qui, au Bureau, président leurs délégations avec engagement- les travaux de certaines de ces délégations auront des conséquences dans cet hémicycle,

l'année prochaine. En application de l'article L.O. 320 du code électoral, le mandat sénatorial de M. Gérard Collomb, dont les fonctions gouvernementales ont pris fin le mercredi 3 octobre 2018,

l'actualité récente nous l'a encore rappelé. L'élection présidentielle brésilienne nous a en effet offert un nouvel exemple de l'utilisation qui peut être faite des réseaux sociaux pour diffuser massivement, et rapidement, de fausses informations. En ce qui concerne les élections de mi-mandat aux États-Unis, qui ont lieu aujourd'hui même, Twitter a supprimé il y a quelques jours des milliers de comptes automatiques qui se présentaient faussement comme démocrates et tweettaient des messages incitant à l'abstention. Cette nuit encore, Facebook a bloqué plus d'une centaine de comptes liés à des entités étrangères et soupçonnés de tentative d'ingérence dans le processus électoral. Partout dans le monde, les fausses informations ébranlent la liberté de chaque citoyen de se forger sa propre opinion. Elles brouillent les frontières entre le vrai et le faux et sapent la confiance dans l'information. Elles menacent, à terme, la stabilité de nos démocraties. Elles nous imposent d'agir. L'Assemblée nationale a choisi de se saisir du sujet au travers de la proposition de loi et de la proposition de loi organique qui nous réunissent aujourd'hui et que le Gouvernement soutient. Je suis convaincu qu'un débat au Sénat en première lecture aurait permis d'enrichir ces textes. Je respecte votre décision de ne pas les avoir examinés en première lecture, mais je la regrette. Je crois en effet que, face à la manipulation de l'information, il serait trop dangereux de ne rien faire. J'ai entendu vos débats, légitimes, autour du référé judiciaire. Son champ d'application a été précisé à l'occasion des lectures successives. Il est très explicitement circonscrit et ne concerne que le contexte particulier de la période électorale. Il vise à nous doter d'outils adaptés pour réagir rapidement à des opérations orchestrées et délibérées de désinformation en période électorale.

Surtout, la lutte contre la manipulation de l'information est un combat au long cours qui ne saurait être remporté grâce à un texte « miracle ». La loi n'est pas la seule réponse que le Gouvernement apporte à cette question. Elle vient en complément de nos actions visant à soutenir la presse, à garantir la déontologie de l'information et à renforcer l'éducation aux médias. La défense et la promotion d'une information pluraliste et de qualité sont nos premières armes pour combattre les tentatives de manipulation de l'information. Je tiens à cet égard à saluer l'initiative lancée par Reporters sans frontières et son secrétaire général, Christophe Deloire, soutenu aujourd'hui par de très nombreuses personnalités, appelant à la signature d'un pacte international sur l'information et la démocratie, première pierre dans l'édification d'un cadre international pour l'information et la communication. Comme l'a indiqué le Président de la République en septembre, la France s'engage à mobiliser l'ensemble des dirigeants internationaux sur ce sujet. Il est en effet de la responsabilité de l'État de garantir le pluralisme de la presse et des médias. Sur ce sujet, la mobilisation du Gouvernement est totale. Les aides au pluralisme sont sanctuarisées à hauteur de 16 millions d'euros dans le budget pour 2019, voté en première lecture la semaine dernière par l'Assemblée nationale. Nous prenons également notre part pour accompagner la mutation de la filière de distribution de la presse, avec la réforme à venir de la loi Bichet- nous aurons l'occasion d'en reparler.

nous continuerons le combat européen pour obtenir la consécration d'un droit voisin. Celui-ci permettra un juste partage de la valeur créée par la circulation en ligne des contenus de presse. Par ailleurs, les débats à l'Assemblée nationale ont fait apparaître un consensus qui dépasse les clivages politiques, autour de la nécessité d'aborder la question de la déontologie de la presse.

La mise en oeuvre de ces propositions concrètes pourra contribuer à restaurer le lien de confiance entre les Français et les médias. Je le répète, les journalistes et la qualité de l'information qu'ils produisent sont à nos yeux le premier rempart contre les fausses informations. L'éducation aux médias constitue également un remède essentiel contre la désinformation. Grâce aux amendements déposés à l'Assemblée nationale, sa place a été renforcée dans la proposition de loi. Elle deviendra un élément obligatoire de l'ensemble des programmes scolaires. En outre, le budget que lui consacre le ministère de la culture a doublé cette année. Il renforcera le soutien des pouvoirs publics aux actions de sensibilisation menées par les professionnels et les associations auprès des jeunes. Il financera aussi la création d'un grand programme de service civique pour l'éducation aux médias. donc la loi n'est pas notre seule arme pour lutter contre la manipulation de l'information, elle est cependant indispensable. Dans le contexte que nous connaissons, il serait dangereux de nous contenter d'attendre une réponse européenne qui tarde encore à venir. Vous le savez, la France a toujours été pionnière en matière de régulation, et nous souhaitons qu'elle le soit encore en matière de régulation numérique. C'est ce que nous encourageons quand nous militons pour la taxation des GAFA ou des GAFAN, quand nous nous battons pour une véritable protection numérique du droit d'auteur ou pour une lutte efficace contre les discours de haine sur internet. le crois, notre responsabilité en matière de lutte contre la manipulation de l'information. Nous avons le devoir de donner l'impulsion, d'expérimenter, d'avancer vers de nouveaux modes de régulation qui pourront permettre d'inspirer ensuite les réponses européennes.

Bien au contraire, elles peuvent y contribuer en proposant des solutions dont l'Union européenne pourrait s'inspirer. Depuis que ces textes ont été annoncés, les instances européennes se sont d'ailleurs emparées du sujet. C'est une bonne chose et je tiens à le saluer. Les initiatives récentes au niveau européen convergent avec l'ambition portée par ces textes. Je pense à la résolution relative à l'affaire Cambridge Analytica, adoptée le 25 octobre par le Parlement européen, ou encore au code de bonnes pratiques publié le 26 septembre dernier par la Commission à l'intention des plateformes internet et des acteurs de la publicité et signé le 16 octobre par Facebook, Google, Twitter et Mozilla. Ces initiatives, si louables soient-elles, ne vont toutefois pas assez loin. Elles ne définissent pas d'engagement suffisamment clair et concret ni d'objectifs mesurables, comme l'ont regretté les professionnels invités à s'exprimer sur le sujet. Surtout, elles ne présentent aucun caractère contraignant pour les plateformes. Or je suis convaincu qu'il serait trop dangereux de s'en remettre uniquement- et même naïvement -, à l'autorégulation des plateformes. Les réseaux sociaux ont récemment pris des mesures afin de lutter contre la diffusion de fausses informations, et c'est tant mieux ! Facebook a, par exemple, renforcé l'information sur les médias d'où proviennent les articles partagés sur son réseau. de ce type démontrent que nous allons dans le bon sens et doivent être encouragées. Les plateformes numériques ont aussi pris conscience de leur responsabilité sociétale et démocratique. Elles reconnaissent de plus en plus clairement l'urgence du combat à mener- une urgence dont elles n'avaient peut-être pas encore pris ou souhaité prendre la mesure il y a encore quelques mois. Elles reconnaissent le bien-fondé de notre exigence d'une transparence renforcée sur les contenus d'information sponsorisés, notamment en période électorale. Les présents textes prévoient de l'inscrire dans la loi. Ainsi, lorsque des techniques publicitaires seront utilisées pour promouvoir un contenu d'information- ce point est très important l'internaute en sera informé et saura d'où provient réellement l'information. Cela contribuera à aiguiser sa vigilance et à mieux le prémunir contre des tentatives de manipulation. De même, les montants consacrés au seront rendus publics. Les journalistes et la société civile pourront mieux détecter les opérations orchestrées de désinformation, et les pouvoirs publics pourront mieux veiller au respect des règles de financement des campagnes électorales. Nous inscrivons également dans la loi un devoir de coopération des plateformes. Cette mesure esquisse un nouveau cadre de régulation adapté à l'ère numérique fondé sur la responsabilisation des plateformes, collectif et transparent, à la fois souple et exigeant. Plutôt que de calquer des mécanismes traditionnels de responsabilité applicables aux médias qui ne leur sont pas pleinement adaptés, les propositions de loi font le choix d'un dispositif de corégulation qui laisse les plateformes libres de choisir les modalités les plus appropriées pour lutter contre les fausses informations, tout en les obligeant à en rendre compte auprès du Conseil supérieur de l'audiovisuel. C'est la seule manière efficace d'éviter les deux écueils qui nous guettent : d'une part, celui de l'inaction des plateformes, qui laisserait la désinformation se propager, troublant la qualité du débat démocratique, voire l'ordre public, et, d'autre et, d'autre part, celui d'une action opaque et arbitraire des plateformes, qui nous ferait courir le risque de l'émergence d'une censure privée. Mesdames les sénatrices, messieurs les sénateurs, ce n'est pas parce que les géants du numérique sont des géants qu'ils peuvent échapper à toute régulation.

Madame la présidente, chère Catherine Morin-Desailly, je connais votre mobilisation sans faille, ainsi que celle de vos collègues de la commission de la culture, et plus largement du Sénat pour que la révolution numérique se fasse au service de nos concitoyens. J'entends aussi vos appels à la prise en main de notre destin numérique. Je n'oublie pas que vous avez été l'une des premières à alerter sur les dangers qu'il pouvait y avoir à confier la gestion de données sensibles à des entreprises qui n'appliquent pas les mêmes règles que nous.

nous permettra de renouer le fil d'un dialogue fructueux au service d'une modernisation de notre régulation. La parole

Madame la présidente, monsieur le président de la commission des lois, monsieur le rapporteur pour avis, mes chers collègues,

de ses fonctions. Mes chers collègues, nous examinons donc aujourd'hui en nouvelle lecture la proposition de loi relative à la lutte contre la manipulation de l'information. Le 26 juillet dernier, par un vote quasi unanime, le Sénat a adopté, sur proposition de sa commission de la culture, une motion tendant à opposer la question préalable à ce texte. Actant un différend irréconciliable, la commission mixte paritaire qui s'est réunie le 26 septembre n'a pas pu trouver un accord. Les députés ont donc examiné en nouvelle lecture la présente proposition de loi le 9 octobre dernier.

Premier point, un large consensus existe aujourd'hui sur la réalité du défi. La proposition de loi traite d'une question qui fait très largement consensus la capacité de certains, en particulier d'États étrangers, à mener des politiques de déstabilisation et de manipulation de l'opinion par le biais des plateformes en ligne. Ce phénomène doit être analysé comme la convergence de deux composantes.

et les mots dépassent souvent la pensée, de notre part comme de celle des militants, ce qui participe par ailleurs de la vitalité démocratique. Il est bien difficile, comme en témoigne une large jurisprudence bâtieautour de la loi de 1881, de faire la part des choses entre liberté d'expression, volonté de nuire ou simple erreur. Les débats à l'Assemblée nationale ont d'ailleurs largement montré que les fausses informations résistent à toute tentative de définition satisfaisante permettant de les identifier rapidement et d'en faire un motif de retrait ou de sanction immédiat. Ce n'est pas la capacité d'une personne à communiquer de fausses informations qui doit être mise en cause, mais bien les modalités de diffusion propres aux plateformes, qui amplifient de manière démesurée ces discours. démesurée ces discours. Ainsi intervient une composante nouvelle, la capacité des réseaux sociaux à amplifier massivement et rapidement des informations, et la possibilité pour certains d'en exploiter les failles. Permettez-moi de citer le remarquable travail du centre d'analyse, de prévision et de stratégie du ministère de l'Europe et des affaires étrangères et de l'institut de recherche stratégique de l'École militaire

et intérêt commercial : « En revanche, il ne faut pas distinguer trop nettement, comme on le fait parfois, les manipulations commerciales dont l'intention serait de faire de l'argent, et qui, pour cette raison, sont souvent dépolitisées par ceux qui les analysent, des manipulations politiques, qui nous intéressent ici. Car non seulement les premières peuvent avoir, qu'elles le veuillent ou non, des effets politiques bien réels, mais les secondes peuvent aussi faire gagner de l'argent aux médias, aux plateformes numériques, voire à des adolescents macédoniens.

au point de ne pas en être discernable, la liberté d'expression, et une réalité nouvelle, car chacun, depuis son ordinateur, ici ou à l'étranger, peutpropager une vision déformée de la réalité pour des motifs politiques ou économiques-souvent les deux.

Fin juillet, Facebook a annoncé avoir détecté une campagne d'influence en cours. Son président a reconnu que la compagnie avait engagé une « course aux armements » avec ceux qui cherchaient à utiliser ses fonctionnalités pour manipuler l'opinion. Il y a quelques jours, vous l'avez rappelé, monsieur le ministre, se tenait l'élection présidentielle au Brésil, qui a été marquée, elle aussi, par la violence des échanges et la polarisation de la société. Le plus remarquable est que le candidat finalement élu ne disposait au départ que d'une très faible notoriété et d'un accès très limité aux grands médias traditionnels. Il a d'ailleurs refusé jusqu'au bout de participer à tout débat télévisé, et a choisi d'axer sa communication sur internet, ce qui lui a permis de tenir des discours destinésà chaque fraction de son électorat

Ainsi, les opinions publiques sont de plus en plus sensibilisées à l'influence des plateformes. On peut faire référence, sur une thématique proche mais pas totalement similaire, au rapport remis au Premier

Par ailleurs, les plateformes elles-mêmes sont désireuses de ne plus prêter le flanc à des polémiques qui nuisent à leur image. Facebook, société la plus fortement accusée de profiter des campagnes de désinformation et, par conséquent, la plus en pointe dans la lutte contre leur diffusion, a inauguré une salle de crise qui va réunir les principaux responsables pour les élections de. Certaines ont signé le code de bonnes pratiques contre la désinformation proposé par Bruxelles et présenté leur plan d'action pour éviter les campagnes de désinformation pendant les élections européennes de 2019. La Commission réalisera une première évaluation en décembre. La commissaire pour l'économie et la société numériques, Mariya Gabriel, insiste sur quatre points : la transparence des publicités politiques sponsorisées, la démonétisation des contenus visant à désinformer, la réduction des faux comptes et des bots, et la promotion des outils à destination des citoyens. Nous ne pouvons que partager pleinement ces objectifs, même s'il

le Sénat de la proposition de loi qui nous est soumise en nouvelle lecture ne signifie nullement que nous refusons de voir la réalité en face. Au contraire, parce que nous savons que ce danger ne disparaîtra pas spontanément et sera présent pendant des années,

En première lecture, conjointement avec Mme la présidente de la commission de la culture, je vous avais proposé, au nom de la commission des lois, de rejeter ces textes, par l'adoption de deux questions préalables. En effet, la création d'une nouvelle procédure de référé, visant à faire cesser la diffusion « des allégations ou imputations inexactes ou trompeuses d'un fait de nature à altérer la sincérité du scrutin à venir », nous paraissait

peut-être naïvement, que l'Assemblée nationale et le Gouvernement cesseraient de s'entêter à vouloir adopter un tel texte et entendraient notre signal d'alerte quant aux risques que font courir la proposition de loi et la proposition de loi organique pour la liberté d'expression et la liberté de communication.

une portée plus opérationnelle »- c'est dire ! -à la définition des fausses informations susceptibles de donner lieu à une procédure de référé. Cette procédure pourrait être engagée lorsque « des allégations ou imputations inexactes ou trompeuses d'un fait de nature à altérer la sincérité du scrutin à venir sont diffusées de manière délibérée, artificielle ou automatisée et massive par le biais d'un service de communication au public en ligne ». Une seconde modification a pour objet de créer une voie d'appel dans le cadre de la procédure de référé instituée pour lutter contre les fausses informations : la cour d'appel se prononcerait dans les quarante-huit heures suivant sa saisine. Ces modifications n'ont pas changé la position de la commission des lois du Sénat : je vous proposerai à nouveau de rejeter les deux textes par l'adoption d'une question préalable.

Je vous rappelle que, durant la campagne pour l'élection présidentielle de 2017, à la suite de la publication des « Macron Leaks », la Commission nationale de contrôle de la campagne électorale en vue de l'élection présidentielle avait demandé aux organes de presse, dans un communiqué de presse daté du 6 mai 2017, de « ne pas rendre compte du contenu de ces données, en rappelant que la diffusion de fausses informations est susceptible de tomber sous le coup de la loi, notamment pénale », puis rappelé, le même jour, que « la diffusion ou la rediffusion de telles données, obtenues frauduleusement, et auxquelles ont pu, selon toute vraisemblance, être mêlées de fausses informations, est susceptible de recevoir une qualification pénale à plusieurs titres et d'engager la responsabilité de ses auteurs. En effet, la publication de fausses nouvelles ayant eu pour effet de fausser un scrutin électoral est déjà réprimée, par l'article L. 97 du code électoral, d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende. Les dispositions actuelles de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse permettent également de réprimer des propos sciemment erronés, diffamatoires, injurieux ou provocants. L'arsenal existe donc. A-t-il été mobilisé ? Pas à ma connaissance. Pourquoi ? Plutôt que d'adapter les dispositions de la loi de 1881 ou celles de la loi pour plutôt que d'en renforcer l'effectivité, le Gouvernement et l'Assemblée nationale ont fait le choix de la création d'un dispositif bancal, intégralement réécrit en première lecture, en commission des lois puis en séance, et à nouveau modifié en nouvelle lecture, ce qui témoigne de ses imperfections structurelles. À l'Assemblée nationale, en première lecture, une première définition de la fausse information a été adoptée en commission, puis en séance, à l'initiative de la rapporteur, ma collègue Naïma Moutchou. Restreint, en commission, aux cas de « mauvaise foi », le recours à la nouvelle voie

puis deux amendements, en séance publique, sur l'initiative de la rapporteur de la commission des lois et du Gouvernement, afin de circonscrire l'application de la procédure de référé, mais également de prévoir une voie d'appel rapide à l'encontre de l'ordonnance de référé, appel devant être jugé dans un délai de quarante-huit heures à compter de la saisine. Alors que la rapporteur souhaitait encadrer la possibilité de faire appel dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la première décision, le Gouvernement a souhaité conserver le délai de droit commun de quinze jours, tout en indiquant se réserver la capacité de modifier, au besoin, ce délai d'appel par décret. Quelle précipitation ! Quelle impréparation pour un sujet aussi sensible ! C'est vrai ! En second lieu, je vous propose de rejeter ces textes, car le dispositif proposé me paraît inefficace contre les vraies menaces. Je ne nie pas les difficultés posées par la diffusion massive de aux fins d'influencer des scrutins : ces manipulations doivent incontestablement être combattues. Mais pourquoi bricoler une loi dans l'urgence sans s'attaquer aux racines des symptômes ? Pourquoi ne pas s'interroger sur les causes profondes du malaise exploité par les ? Pourquoi le complotisme séduit-il ? Pourquoi une telle défiance envers les élites politiques ou intellectuelles ? Je ne suis pas sûr qu'une nouvelle procédure répressive, réclamée par le Président de la République et le Gouvernement, soit la réponse la plus efficace à ces mouvements qui tentent de décrédibiliser la parole publique. Les vraies manipulations de l'information sont délibérées, mais surtout clandestines : elles ne sont évidentes ni pour le public ni pour les victimes de ces manipulations. Elles ne peuvent donc être appréhendées par un dispositif judiciaire exigeant de rapporter la preuve contraire et des allégations proférées. Je rappelle que le juge des référés est le juge de l'évidence, de l'illégalité manifeste. En quarante-huit heures, il ne peut, en principe, statuer que sur des mensonges évidents ou manifestes. Toutefois, peut-on encore considérer qu'il y a tromperie des électeurs en cas d'allégation manifestement erronée ou outrancière ? Monsieur le ministre, vous avez déclaré qu'il s'agissait d'« un premier pas vers une meilleure responsabilisation des plateformes numériques. » Vous savez très bien que c'est erroné ! Seule une législation européenne pourrait permettre une responsabilisation accrue des plateformes numériques. Ce choix d'un dispositif franco-français est un choix d'inefficacité contre les vraies manipulations de l'information menées par des acteurs étrangers, qui resteraient à l'abri de ces dispositions. Il est regrettable que, pour un dispositif inefficace contre les vraies menaces, le Gouvernement et l'Assemblée nationale soient prêts à remettre en cause la tradition française de liberté d'expression en matière politique. en troisième lieu, de rejeter ces textes, qui, tout en étant inefficaces contre les vraies menaces, pourraient être instrumentalisés au détriment de la liberté d'expression. Je rappelle que, contrairement à ce que prétend le Gouvernement, qui affirme que la procédure de référé sera limitée aux seules

sera concernée toute allégation, même satirique, même parodique, « de nature » à altérer la sincérité d'un scrutin à venir et non les seules allégations diffusées avec une intention malveillante ou délibérée d'altérer la sincérité d'un scrutin à venir. Qu'une allégation soit « de nature » à altérer un scrutin ne signifie pas qu'elle ait été diffusée avec cette intention ! Le texte adopté par l'Assemblée nationale permet à n'importe qui de saisir le juge des référés. C'est une porte ouverte aux instrumentalisations. L'autorité judiciaire est incontestablement la gardienne des libertés individuelles, notamment de la liberté d'expression. Mais aucun juge n'est infaillible, lorsque la loi l'oblige à statuer en Comment le juge des référés pourrait-il, en quarante-huit heures, établir l'altération d'un scrutin qui n'a pas eu lieu ? Une telle législation risque d'engendrer des décisions contestables, au risque, d'ailleurs, de jurisprudences contraires entre le juge judiciaire et le juge de l'élection, donc un affaiblissement de notre justice. La sincérité des scrutins risquerait, elle aussi, d'être affaiblie en cas de décision d'appel contredisant le juge des référés de première instance, notifiée après le scrutin. Le juge de l'élection serait-il tenu par cette décision ? Quelle légitimité pour les gagnants d'une élection ? Outre le risque d'affaiblir la liberté d'expression, ces dispositions présentent bien un danger démocratique. Mes chers collègues, puisque le Sénat est attaché aux libertés fondamentales, je vous proposerai, une fois encore, d'adopter une motion tendant à opposer la question préalable sur la proposition de loi organique. Nous passons Nous passons à la discussion de la motion tendant à opposer l'exception d'irrecevabilité sur la proposition de loi.

qui proclame que « La libre communication des pensées et des opinions est un des droits les plus précieux de l'homme : tout citoyen peut donc parler, écrire, imprimer librement, sauf à répondre de l'abus de cette liberté dans les cas déterminés par la loi.

ce qui ne nuit pas à autrui ». En d'autres termes, la liberté d'opinion et la liberté d'expression sont intrinsèquement fondées sur une éthique de responsabilité. L'ensemble de notre droit positif interne repose sur cet équilibre entre reconnaissance, consécration de la liberté d'expression et répression de ses abus.

s'avèrent constituer une entrave manifeste et disproportionnée à la liberté d'expression et à la liberté d'information. Il convient de rappeler ici que le Conseil constitutionnel a souligné, selon une jurisprudence constante, que « la liberté d'expression et de communication est d'autant plus précieuse que son exercice est une condition de la démocratie et l'une des garanties du respect des autres droits et libertés. » Par conséquent, elle est une forme de droit premier, à la fois individuel et collectif, qui conditionne la nature d'un régime politique, caractérise son degré démocratique et assure l'effectivité d'autres droits dérivés ou, tout du moins, de droits dont l'exercice dépend de celui de la liberté d'expression et de communication, à l'image, par exemple, de la liberté de la presse. Elle est donc un droit éminemment ordonnateur. présent texte est porteur, en lui-même, d'un risque de censure, qui menace la liberté d'expression, d'information et de la presse, d'autant plus que la notion de « fausse information » n'est même plus explicitée. Certes, la définition qui figurait initialement dans le texte était imparfaite, mais l'avoir purement et simplement effacée était-elle vraiment la solution ? Pour résumer, nous nous retrouvons à légiférer sur un sujet important, sans même avoir pris le temps de le définir clairement. Dans ce contexte, comment pouvons-nous établir des dispositifs législatifs pertinents ou caractériser clairement des infractions pénales ? Le risque est d'ouvrir la boîte de Pandore et d'offrir inutilement des instruments à ceux qui pourraient être tentés de les utiliser à des fins hautement pernicieuses,

les solutions apportées sont constitutionnellement chancelantes à l'égard du droit fondamental que constitue la liberté d'expression et de communication. Par ailleurs, ce texte paraît porter atteinte aux principes constitutionnels de la liberté du commerce et de l'industrie ainsi que de la liberté d'entreprendre, pour des motifs divers. tout d'abord, à l'obligation de transparence imposée aux plateformes en période d'élections. Dans son avis, le Conseil d'État a mis en exergue que seul le rattachement de cette obligation à une « raison impérieuse d'intérêt général inédite », s'attachant à préserver l'information éclairée des citoyens en périodes électorales », était de nature à la justifier. Si les députés ont effectivement pris le soin d'introduire cette précision, l'absence de définition de la notion d'« information éclairée » ne motive aucunement l'application de cette obligation, que la Cour de justice de l'Union européenne, la CJUE, a déjà condamnée à plusieurs reprises. Je pense, ensuite, à la situation de concurrence déloyale induite dès lors que certains médias peuvent se retrouver privés d'une exposition « juste et équitable Ce pourrait être le cas pour les sites ou les pages supprimés à la suite de l'intervention du juge des référés, conformément à l'article 1, pour les services audiovisuels qui verraient leur convention unilatéralement résiliée par le Conseil supérieur de l'audiovisuel, le CSA, même hors période électorale, en vertu de l'article 6, ou leur distribution ou diffusion suspendues par cette instance pendant la période électorale.

Autrement dit, la mise en oeuvre des articles du titre II entraînerait une rupture d'égalité manifeste en termes de libre concurrence, autre principe constitutionnel sur lequel l'Union européenne et la CJUE sont très vigilantes. De plus, la faculté de résiliation unilatérale de la convention par le CSA, ouverte par l'article 6 de la proposition de loi, interroge fortement. Le Conseil constitutionnel, dans sa décision du 10 juin 2009 sur la loi favorisant la diffusion et la protection de la création sur internet, a censuré des dispositions qui visaient à conférer à une autorité administrative indépendante, ou AAI, des pouvoirs de sanction inadaptés et excessifs. Postulant qu'une AAI « n'est pas une juridiction », que les pouvoirs de sanction octroyés par le projet de loi « peuvent conduire à restreindre » le « droit de s'exprimer et de communiquer librement », le Conseil conclut que, « eu égard à la nature de la liberté garantie par l'article XI de la Déclaration de 1789, le législateur ne pouvait, quelles que soient les garanties encadrant le prononcé des sanctions, confier de tels pouvoirs à une autorité administrative

que « le fait de sanctionner une personne morale en raison des seuls agissements commis par d'autres personnes morales, qui peuvent être sans lien direct avec elle », ce qui serait le cas, par exemple, des filiales de l'actionnaire de la société, « apparaît difficilement conciliable avec les principes constitutionnels de responsabilité personnelle et de personnalité des peines, garantis par les articles VIII et IX de la Déclaration de 1789 ». Enfin, d'autres points juridiquement douteux et singulièrement flous laissent à penser que nous devons, en tant que législateurs, preuve d'incompétence négative. En effet, le Conseil constitutionnel est « attentif à ce que le législateur ne reporte pas sur une autorité administrative [ ...] ou sur une autorité juridictionnelle le soin de fixer des règles ou des principes dont la détermination n'a été confiée qu'à la loi », en vertu de l'article 34 de la Constitution. À cet égard, ce dernier a été élargi au secteur des médias lors de la réforme constitutionnelle de 2008, que vous connaissez bien, monsieur le ministre, grâce à un amendement des sénateurs socialistes. Désormais, le législateur a compétence pour établir les règles concernant « la liberté, le pluralisme et l'indépendance des médias Par ailleurs, l'incompétence négative est caractérisée quand « le législateur élabore une loi trop imprécise ou ambiguë » ou qu'il renvoie au pouvoir réglementaire « de façon trop générale ou imprécise ». Or, comme cela a été démontré précédemment, le coeur même de ce texte, à savoir « la fausse information », n'est nullement défini. Aussi, étant donné cette imprécision générale et constante, de nombreux contentieux risquent d'éclore et quantité d'inconnues demeurent. Comment le juge des référés pourrait-il se prononcer sur des faits de nature à influencer un scrutin encore non advenu ? Comment effectuer un contrôle sur un événement dont l'aboutissement est, par nature, incertain ? Que signifie un service audiovisuel « sous influence » d'un État étranger ? En l'état, cette notion juridique est inexistante dans notre droit positif. Il eût été primordial de l'encadrer et de déterminer des critères qui permettent de l'appréhender. En conclusion,

Quel est l'avis de la commission ?

des journalistes, malgré les dangers pour la liberté d'expression, malgré l'inutilité et l'inefficacité des dispositions prévues, sur le plan politique comme sur le la discussion du texte n'a laissé place à aucun travail transpartisan, ni à aucune recherche d'un consensus minimal entre les partis démocratiques et républicains. D'ailleurs, dans les deux assemblées, seuls les partis de la majorité l'ont voté.

le 26 septembre dernier, sénateurs et députés réunis en commission mixte paritaire ont fait le constat d'un différend irréconciliable sur les textes relatifs à la lutte contre la manipulation de l'information.

Les observations que nous avions formulées s'inscrivaient pourtant dans une démarche réellement constructive. Il n'y avait et il n'y a toujours de notre part aucune forme d'obstruction politique à la démarche engagée par la majorité gouvernementale. Personne ne nie l'importance de préserver le débat public des fausses informations. Nous sommes convaincus qu'elles appellent de notre part une réflexion approfondie.

Cela illustre le consensus qui existe parmi nous sur ce sujet, comme sur l'analyse que nous voulons en faire. Nous sommes toutes et tous convaincus de la nécessité d'agir. à ce qui a pu être affirmé à l'Assemblée nationale, nous n'estimons pas nécessairement que, « en matière de lutte contre les fausses informations, notre arsenal juridique est suffisant ni qu'aucune évolution des textes existants n'est souhaitable. Nous ne jugeons pas non plus préférable « de laisser aux seules plateformes le soin de réguler l'information Enfin, nous ne considérons pas que « l'éducation aux médias, en particulier pour les plus jeunes, n'est pas un enjeu central et primordial du combat que nous voulons mener La réalité est tout autre : nous ne nous retrouvons pas dans les propositions qui nous sont faites par nos collègues députés membres de la majorité. À la vérité, les fondements mêmes de ce texte ne conviennent pas.

S'il y a flagrance, son action sera en quelque sorte inutile. En l'absence de flagrance, si le juge, par prudence, décide de ne pas se prononcer, il légitimera d'une certaine façon l'information diffusée.

Quant aux dispositions relatives à la formation au numérique et aux médias, notamment des plus jeunes, elles sont souhaitées et souhaitables, mais force est de constater que celles qui ont déjà été introduites par le Sénat en 2011 n'ont toujours pas trouvé de cadre d'action global. Les sénateurs du groupe du RDSE se félicitent tout de même de l'annonce- même si elle ne s'inscrit pas dans le cadre législatif dont nous débattons cet après-midi -du lancement d'une mission confiée à l'ancien président de l'Agence France Presse et visant à créer une autorité de déontologie de la presse. En effet, l'un des remparts les plus efficaces contre la désinformation et la manipulation de l'information demeure les médias et ceux qui les animent, les journalistes. Pour l'avenir, employons-nous à travailler en harmonie avec l'Union européenne. C'est à ce niveau que, dans un souci d'efficacité et de respect des libertés fondamentales, le combat est à mener. Pourquoi créer une procédure spécifique à l'échelle nationale, alors que, même si l'on peut estimer qu'ils évoluent encore trop lentement, les travaux européens sur le sujet avancent et tendent à établir une régulation plus générale ?

Notre abstention vise à rappeler que, si notre groupe, avant tout favorable au débat, ne s'associe habituellement pas aux motions de procédure, il est pleinement conscient que, pour reprendre les mots du président Bas, ces deux textes ne sont pas « améliorables je vous remercie

Ce que l'on appelait autrefois, dans l'ancien monde, quand la France était francophone, les racontars, cela a toujours existé. Récemment encore, ces racontars n'ont pas empêché Emmanuel Macron d'être élu Président de la République. À moins qu'ils ne le lui aient permis- vous voyez, mes chers collègues, que, à force de voir des partout, on finirait presque par douter de la sincérité des urnes ... La réalité, quelle est-elle ? Une étude conjointe du CNRS et de l'École des hautes études en sciences sociales révèle que, sur 6 millions de tweets analysés, eux seulement comporte un lien référencé comme une fausse information. De toute évidence, il y a davantage de rumeurs et de manipulations dans et dans, pour ne citer qu'eux, que sur les réseaux sociaux À vrai dire, il n'y a pas de fumée sans feu. Si certains répandent de fausses informations, c'est peut-être que les politiques hésitantes, mais toujours contraignantes du Gouvernement déboussolent nos compatriotes, qui n'accèdent pas à l'esprit complexe, pour ne pas dire tourmenté, d'Emmanuel Macron, et que, forts de ce constat, certains sont tentés de penser que la vérité est ailleurs. Ce texte participe d'un climat délétère de dérives liberticides d'un pouvoir qui, après seulement dix-huit mois d'exercice, est déjà à l'agonie. On ferme les réseaux sociaux des militants politiques qui ne pensent pas comme il faut, contre toute règle de droit. Vexations, intimidations et mises en examen sont largement relayées par le tribunal médiatique, dont certains organes n'ont rien à refuser au locataire de l'Élysée. De Fillon à Mélenchon, en passant par Marine Le Pen et le Rassemblement national, on persécute les partis politiques d'opposition.

En réalité, vous cassez le droit en vigueur. Finie la justification d'un fait précis : ce texte permettra de supprimer des contenus de manière aléatoire. C'est ce qu'on appelle museler l'information, effectivement, cela sent curieusement les années trente ! Ce texte vague et largement interprétable n'est pas acceptable. Il représente un danger pour nos libertés institutionnelles, pour les libertés individuelles, et,, pour la démocratie. Je crains que l'on ait pris l'habitude de vouloir museler le peuple et son droit à défendre ses aspirations profondes, aujourd'hui sa volonté de tourner la page du prétendu nouveau monde- le plus grand politique des dix dernières années pourtant légitime que le peuple aspire à un réel changement, quand vous vous contentez de coups de com'pour tenter de sauver l'ultralibéralisme et l'impérialisme de Bruxelles. Qu'il me soit permis de dénoncer cette lancée en son temps par François Mitterrand et reprise aujourd'hui par l'actuel Président de la République : non, le nationalisme, ce n'est pas la guerre

aux débats de fond et, plutôt que d'empêcher, de fermer et de supprimer, libérons et confrontons la diversité d'opinions, terreau indispensable à la liberté démocratique

Madame la présidente, monsieur le ministre, madame la présidente et rapporteur de la commission de la culture, monsieur le rapporteur de la commission des lois, mes chers collègues, lors des dernières élections présidentielles au Brésil, 100 000 comptes WhatsApp ont inondé la plateforme de centaines de millions de messages de soutien à la campagne de Jair Bolsonaro. Cette pratique, pour être tout à fait illégale, n'en est pas moins efficace.

Ensuite, la tentative d'ingérence dans l'élection présidentielle française de 2017 nous a fait prendre conscience plus concrètement de notre vulnérabilité. La manipulation de l'information, entendue comme la diffusion intentionnelle et massive de nouvelles fausses ou biaisées à des fins politiques hostiles, est liée à la combinaison de deux facteurs : d'une part, les capacités de diffusion rapide offertes par internet et les réseaux sociaux ; d'autre part, la crise de confiance qui dévalue la parole publique « Une idée fausse, mais claire et précise, aura toujours plus de puissance dans le monde qu'une idée vraie, mais complexe », disait Alexis de Tocqueville, à l'époque où les fausses informations circulaient encore à la vitesse des machines à vapeur. La généralisation des réseaux sociaux et des pratiques de change la donne : un quart de seconde suffit désormais pour qu'une théorie complotiste franchisse l'Atlantique, et en quelques heures seulement, avec quelques milliers d'euros, une campagne de désinformation politique peut devenir virale. Pour contrer ce phénomène, l'Assemblée nationale nous transmet une seconde fois une proposition de loi visant à lutter contre la manipulation de l'information en période électorale. Nous savons tous qu'il est nécessaire d'agir pour protéger nos démocraties. Une première fois, le 26 juillet dernier, le Sénat a fait le choix de ne pas examiner ce texte, au lieu de l'amender et d'en proposer une réécriture en vue d'une conciliation en commission mixte paritaire. Notre groupe s'était opposé à cette décision, jugeant que la Haute Assemblée devait exercer sa responsabilité législative. Nous maintenons notre position. Si les lois actuelles étaient suffisantes pour résoudre le problème de la désinformation en période électorale,

Les modes de diffusion étaient alors radicalement différents, sans audiovisuel, sans réseaux sociaux ni plateformes numériques. La régulation des plateformes est un volet essentiel du texte. Il ne s'agit pas de confier aux géants du web la privatisation de nos libertés, mais de retirer le plus rapidement possible des contenus illégaux qui risqueraient de déstabiliser un candidat et de changer le cours d'une élection, voire de l'Histoire. Les GAFA ont leur part de responsabilité dans la diffusion de tels contenus : nous devons les inviter à coopérer, et c'est précisément ce que prévoit la proposition de loi. À l'heure où 83 % des jeunes s'informent sur internet, notamment sur les réseaux sociaux, je ne pense pas qu'il soit judicieux de se cacher derrière le droit européen, qui a sa propre force d'inertie, et d'attendre qu'il évolue. Pour autant, nous reconnaissons la modestie de cette proposition de loi, qui ne permettra pas la disparition complète des fausses informations d'ailleurs plutôt une bonne nouvelle, car un dispositif d'une telle efficacité serait dangereux pour les libertés individuelles. L'information est un enjeu et un instrument de pouvoir. Sa manipulation est un venin pour notre démocratie : elle mine de l'intérieur la confiance des citoyens envers leurs représentants.

Il nous semble que la contribution de la chambre haute du Parlement est d'autant plus importante que le sujet est éminemment politique et sensible ! La parole

Par ailleurs, monsieur le ministre, vous avez récemment confirmé la mise en place prochaine, en complément de cette proposition de loi, d'un Conseil de la déontologie de l'information, où journalistes et éditeurs seront largement représentés. Cette instance, que que nous avons maintes fois appelée de nos voeux et qui existe déjà dans dix-huit pays de l'Union européenne, sera très utile. Il ne s'agira nullement d'un tribunal de la pensée ou d'une instance de censure, ainsi que certains se plaisent déjà à la décrire. Elle émettra

de loi. Ses avis permettront notamment d'éclairer et de légitimer les décisions que le juge des référés sera amené à prendre.

L'opposition au Gouvernement parle d'un texte bâclé, d'une proposition mal ficelée et même d'une législation qui serait dangereuse pour nos libertés, en particulier pour la liberté d'expression.

Ainsi, sont évoquées de « vraies manipulations de l'information », de « vraies entreprises de manipulation » et, par deux fois, de « vraies menaces

Je pense pouvoir entendre tous les arguments, mais je me méfie toujours de celles et de ceux qui, en guise d'argument définitif, prétendent détenir la vérité, la seule vérité. Mes chers collègues, j'ai bien peur que nous soyons au coeur de ce que Guy Debord résumait par cet aphorisme : « Dans un monde réellement renversé, le vrai est un moment du faux Notre monde réel n'est heureusement pas encore totalement renversé, mais l'actualité récente, qu'il s'agisse de l'élection présidentielle au Brésil ou de la campagne de mi-mandat aux États-Unis, nous montre que, d'ores et déjà, le faux est devenu un moment du vrai.

: où sont passés les législateurs que nous sommes pendant tout ce temps ? Renvoyer la solution au problème de la prolifération inquiétante des fausses nouvelles à un renforcement de l'éducation aux médias relève de l'esquive, pour ne pas dire de l'escamotage. D'autant que celles et ceux qui le prônent ici ne se sont pas toujours mobilisés quand les moyens publics alloués à cette entreprise ont décliné durant la décennie écoulée. De même, prôner l'autorégulation, rien que l'autorégulation, par les médias eux-mêmes est une manière assez sournoise de laisser la situation se dégrader encore et encore. En effet, nous avons plus affaire non plus à des médias déclarés responsables de la qualité et de la crédibilité des informations qu'ils délivrent, mais à une de plateformes sans frontières, qui propagent massivement des flux d'informations dont elles ne sont ni les productrices ni les garantes de la valeur informative. La réalité grandissante d'aujourd'hui, c'est que l'on s'informe de moins en moins, mais que l'on est de plus en plus informé, c'est-à-dire soumis à des flux d'informations

Madame la présidente, monsieur le ministre, mes chers collègues, le Président de la République, à l'occasion de ses voeux à la presse du 3 janvier dernier, a demandé une loi sur les fausses informations avant la fin de l'année. Le Gouvernement a jugé que satisfaire cette exigence lui imposait d'en passer par une proposition de loi, dans le cadre de la procédure accélérée, qui lui permettrait d'aller vite et, partant, d'échapper à une évaluation scrupuleuse des conséquences Il y a toujours péril à intervenir par la loi sur des matières touchant aux fondements de notre démocratie, comme la liberté de l'information, surtout de façon aussi expéditive. En l'espèce, les craintes nombreuses et légitimes exprimées par différents acteurs auraient dû amener le Gouvernement à plus de concertation, d'attention et de circonspection. Las, insensible aux réserves et craintes exprimées, vous avez demandé au groupe majoritaire de l'Assemblée nationale, bien docile, de tenter de parachever une proposition de loi d'initiative présidentielle que votre prédécesseur elle-même jugeait très perfectible.

Sans rien écouter des réserves de fond émises à l'intérieur comme à l'extérieur du Parlement, votre gouvernement a décidé de poursuivre l'examen de ce texte, à la hussarde.

de ses commissions, suivies par un hémicycle quasi unanime, d'opposer à votre texte la question préalable. Le Sénat l'a fait en pleine conscience de ses responsabilités particulières en faveur de la défense des libertés démocratiques et individuelles et en expliquant dans le détail pourquoi les dispositions de ce texte étaient au mieux inopérantes, au pire liberticides. C'est donc avec un sentiment mêlant l'injustice à l'improbité que nous recevons les propos fort peu amènes de la rapporteur de la commission des lois de l'Assemblée nationale, qui considère que le Sénat n'a pas « joué le jeu », a fait « un choix politique », un « choix de posture » et a rejeté le texte « sans aucun argument fondé ». Je regrette qu'elle n'ait pas lu l'argumentaire produit par une très large majorité de cet hémicycle. L'eût-elle fait qu'elle aurait paradoxalement constaté que certains des arguments avancés par notre chambre haute avaient été repris,, par le rapporteur de la commission des affaires culturelles de l'Assemblée nationale. Ainsi, ce dernier reconnaît notamment que la loi du 29 juillet 1881 « répond assez largement au problème des fausses informations l'article 27 de cette loi prévoit que « la publication, la diffusion ou la reproduction, par quelque moyen que ce soit, de nouvelles fausses, de pièces fabriquées, falsifiées ou mensongèrement attribuées à des tiers lorsque, faite de mauvaise foi, elle aura troublé la paix publique, ou aura été susceptible de la troubler, sera punie d'une amende de 45 000 euros ». Vous avez choisi, avec la présente proposition de loi, de traiter les « fausses informations », quand la loi de 1881 réprime les « nouvelles fausses La place de l'adjectif, avant ou après le nom, a de la valeur en français. En l'occurrence, elle explicite clairement l'intention du législateur de 1881, qui a retenu, pour que l'infraction soit constituée, le critère fondamental de l'intentionnalité il n'y a d'informations fausses que lorsque les faits ont été manipulés à dessein pour nuire, alors que la fausse information peut être diffusée sans volonté de falsification. Dans son avis du 19 avril dernier, le Conseil d'État vous avait mis en garde contre l'imprécision de l'expression « fausse information ». Il avait recommandé que « la lutte contre les fausses informations soit systématiquement circonscrite aux cas dans lesquels il est établi que la diffusion de telles informations procède d'une intention délibérée de nuire ». Vous avez décidé de ne pas suivre sa recommandation. Peut-être avez-vous jugé qu'il s'agissait aussi d'un choix de posture ans après sa promulgation, la loi de 1881 est toujours opérante, car elle a su trouver un compromis satisfaisant entre la défense de la liberté d'opinion et la lutte contre la diffamation. Pourquoi est-elle alors d'une efficacité peu probante pour endiguer le flux des calomnies et des accusations malveillantes déversées par les plateformes des réseaux sociaux ? Précisément parce que ces dernières refusent d'être assimilées à ces organes de publication, de diffusion ou de reproduction visés par la loi précitée. Tant que ces plateformes refuseront absolument toutes les responsabilités qui incombent à l'éditeur en arguant qu'elles ne font que mettre en relation des lecteurs et des producteurs de données, il n'y aura pas de solution légale pour tenter de réglementer leurs activités. Vous le reconnaissez vous-même, monsieur le ministre, en tentant d'obtenir de ces plateformes le respect, non contraignant, de règles de bonne conduite. Comment croire qu'elles les respecteront, alors que leur modèle économique leur impose de se placer au-dessus des lois ?

le 26 juillet dernier, je précisais à cette même place, au nom du groupe Union Centriste, précisant qu'il n'y avait pas lieu de poursuivre la discussion en séance publique de cette proposition de loi, tant celle-ci apparaissait à la fois inutile et dangereuse, une position d'ailleurs partagée par la très grande majorité des professionnels auditionnés à l'occasion de l'analyse de ce texte. Aujourd'hui, force est de constater que rien n'a changé ... ou si peu. La commission mixte paritaire n'a proposé aucune avancée significative. Permettez-moi, dans un premier temps, de citer un récent rapport établi par le Centre d'analyse, de prévision et de stratégie et l'Institut de recherche stratégique de l'École militaire, qui souligne notamment : « Les manipulations de l'information ne sont pas un phénomène nouveau. Leur actualité récente est liée à la combinaison de deux facteurs : d'une part, les capacités inédites de diffusion rapide et de viralité offertes par internet et les réseaux sociaux, couplées, d'autre part, à la crise de confiance que vivent nos démocraties et qui dévalue la parole publique, allant jusqu'à relativiser la notion même de vérité. » Comme précisé en juillet dernier, à l'heure d'internet et des réseaux sociaux, la question de la manipulation de l'information est, certes, un sujet majeur, mais les dispositions du présent texte ne sont pas de nature à y répondre de manière satisfaisante. Ce rapport précise en outre : « Les élections américaines de 2016 et françaises de 2017 ont jeté une lumière crue sur ce phénomène, ses ressorts et ses conséquences. » Il pose la question suivante : « Ne sommes-nous pas dans le cadre du débat démocratique, dont les excès peuvent être corrigés par la législation en vigueur ?

Le chapitre IV de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse porte expressément sur « les crimes et délits commis par la voie de la presse ou par tout autre moyen de publication ». La création d'un nouveau dispositif ne se justifie donc pas. De plus, la viralité des réseaux sociaux rendra inopérantes les sanctions prévues par le texte. En effet, que vaut le retrait d'un contenu par une plateforme s'il a pu être dupliqué à des milliers ou des millions d'exemplaires par les utilisateurs en quelques secondes ? l'audiovisuel, le CSA, sont investis de missions qu'ils ne pourront pas remplir. La notion de « manipulation de l'information » est très vague, et le texte ne parvient pas à l'expliciter de manière satisfaisante. Le juge aura du mal à disposer des éléments qui lui permettront de se prononcer sous quarante-huit heures. Il se déclarera sans doute souvent incompétent. Comment affirmer qu'un juge des référés pourra établir qu'une « fausse information » est de nature à altérer la sincérité d'un scrutin, qui, par définition, n'a pas encore eu lieu ? De même, qu'est-ce qu'une chaîne « contrôlée » ou « sous l'influence » d'un État étranger ? Le CSA se retrouvera, donc, dans la même situation que le juge des référés. Par certains aspects, le texte peut même apparaître dangereux. Dangereux, pour la liberté d'expression. Sous couvert de lutte contre la manipulation de l'information, le dispositif ne permettra-t-il pas d'étouffer certaines affaires ? Dangereux, parce qu'il est générateur de discriminations : oui, le texte crée une discrimination entre le monde politique et le reste de la société. En effet, la question de la manipulation de l'information se pose à tous les citoyens. Or ce texte peut apparaître comme une réponse corporatiste, destinée simplement à protéger le monde politique. Il aurait vocation à ne s'appliquer qu'à l'occasion des campagnes électorales pour protéger les candidats. Il s'agit donc d'un texte de protection des élus, voté par des élus. élus. de la manipulation de l'information dont peuvent être victimes quotidiennement nos concitoyens ? De plus, le texte semble créer une discrimination entre les journalistes dont les médias ont une édition « print » et les journalistes dont les médias sont dits « pure player ». Seuls ces derniers, alors qu'ils sont des journalistes à part entière, seraient soumis au dispositif prévu par le texte. Pour toutes ces raisons, la présente proposition de loi apparaît comme un texte épidermique,

Ce n'est pas à notre niveau que cette question doit être traitée ; il faut l'appréhender au niveau européen. C'est pour cette raison que la proposition de résolution européenne déposée par la présidente de la commission de la culture, Mme Catherine Morin-Desailly, sur la responsabilisation partielle des hébergeurs va dans le bon sens, celui d'un cadre européen unifié. unifié. Monsieur le ministre, je le rappelle une nouvelle fois, la meilleure des choses pour lutter contre les fausses informations serait de permettre la diffusion de la véritable information. Pour ce faire, il est temps d'assurer, enfin, une parfaite distribution de nos journaux et magazines de presse écrite sur l'ensemble du territoire, en faisant évoluer la loi Bichet, mais j'ai entendu que vous y étiez tout à fait sensible. Pour conclure, je ne comprends toujours pas cet entêtement à vanter les mérites d'un texte fait à la hâte, qui ne répond à aucune priorité étatique et qui, je le réaffirme, est inégalitaire, injuste, discriminatoire et dangereux. C'est pourquoi nous voterons bien sûr les deux motions. La

qui sont tout à fait mobilisables, telles que le référé de droit commun ou les procédures d'injure ou de diffamation entre autres. La réforme envisagée se traduit principalement par deux types de mesures : d'une part, une nouvelle action en référé, qui met en danger la liberté d'expression dans les campagnes électorales, et, d'autre part, une régulation franco-française des plateformes, alors que celle-ci devrait s'élaborer au niveau européen. Notre position est bien claire : nous sommes pleinement conscients de la nécessité de lutter contre les fausses informations, mais nous ne cautionnons ni l'orientation ni les choix que porte ce texte adopté par l'Assemblée nationale, appuyé par le Gouvernement. La difficulté de caractériser la « fausse information » est apparue dès le départ à l'Assemblée nationale, qui, contrainte d'honorer la promesse du Président de la République, a beaucoup souffert pour en donner une définition. Les rédactions successives ont bien montré l'impréparation de ce texte et les hésitations liées aux risques d'atteinte à la liberté d'expression. Finalement, aucune intention malveillante n'est exigée, ce qui ouvre un large champ d'application. Même les actes de satire ou de parodie, voire de caricature, inhérents à l'expression de notre pays, pourraient être concernés. N'importe quel courant de pensée pourra tenter d'empêcher la publication d'informations dérangeantes, alors même qu'il est légitime pour le citoyen d'être informé, surtout, précisément en période électorale. Une vraie information pourra être arrêtée par manque de preuves ou impossibilité de citer ses sources. Les exemples de scandales politiques qui auraient pu être traités comme des à leur origine ailleurs, l'absence de condamnation du juge, faute de preuves ou de moyens d'investigation, pourra donner une force imprévue aux allégations en cause, qui pourront continuer à être diffusées. De quels moyens le juge disposera-t-il pour rendre son verdict en quarante-huit heures ? Comment pourra-t-il affirmer l'influence d'informations sur un scrutin qui n'aura pas encore eu lieu, et son intervention ne risque-t-elle pas d'être remise en cause par la suite ? Le remède risque d'être pire que le mal. On aboutira finalement, quelle que soit l'issue de la procédure judiciaire, à une publicité supplémentaire, ce qui n'est pas le but et ne satisfait personne. Les autres instruments prévus ne sont guère plus solides. L'extension des pouvoirs du CSA et la régulation du numérique sont décidées sans aucune concertation préalable. Finalement, le Gouvernement demande aux juges, au CSA et aux plateformes d'être les gardiens de la vérité.

Le sujet est actuellement étudié au niveau européen, comme cela a été dit. La Commission européenne vient de publier un code de bonne conduite, qui donnera lieu à une évaluation en décembre prochain. La dimension transfrontalière de la désinformation en ligne est évidente et rend nécessaire cette approche. Notre groupe regrette donc la précipitation du Gouvernement, qui place notre pays dans une logique de contrôle de l'information, que nous refusons d'entériner.

Monsieur le rapporteur, vous faites une mauvaise interprétation de l'article 1. Le juge des référés ne pourra ordonner la suspension qu'en cas de diffusion massive, artificielle et délibérée d'une nouvelle

inadmissibles. Dès ma prise de fonctions, j'ai réaffirmé la nécessité de protéger les journalistes, ainsi que la liberté et le pluralisme de la presse ; c'est fondamental. Je me suis exprimé devant le Syndicat national des journalistes, pour dire que je serai toujours

Alors que se terminent les commémorations du centenaire de la Grande Guerre, qui ont permis pendant plus de quatre ans de nous rappeler l'horreur de la guerre, les sacrifices de nos aînés,

de numérisation des archives, notamment des matricules des poilus. Plus de 9,5 millions de matricules ont été numérisés par les archives départementales, en lien avec les Archives nationales. Un portail national a été créé, le grand mémorial des poilus, qui permet

lois. Monsieur le ministre, j'ai écouté avec attention votre réponse aux différents orateurs. Vous avez notamment estimé que nous serions en

Ce ne sont pas simplement les fausses informations qu'il faut traquer, mais aussi ceux qui les diffusent, les fabriquent et les répandent. Cette législation est dangereuse, parce qu'il s'agit

est également inaboutie. En témoignent d'ailleurs les variations que ce texte a subies pendant toute sa préparation et les hésitations dont il a été assorti.

la distinction entre le faux et le vrai n'est pas si nette dans le débat politique, puisqu'elle est en réalité l'expression d'opinions divergentes.

Mme la rapporteur, pour la motion. Madame la présidente, monsieur le ministre, mes très chers collègues, il me revient de défendre devant vous, pour la seconde fois sur ce texte, la motion tendant à opposer la question préalable. Tout d'abord, je veux très solennellement rappeler que le choix de ne pas entamer le débat n'est pas inscrit dans l'ADN du Sénat. C'est vrai ! Nous préférons toujours engager un dialogue avec le Gouvernement et la majorité de l'Assemblée nationale, quelle qu'elle soit, pour faire avancer nos idées, celles qui sont chères à notre assemblée,

en première lecture, au nom de la commission de la culture, a été adoptée par 288 voix contre 31. On sait bien, monsieur le ministre, les conditions dans lesquelles

Mal calibrée, celle-ci n'aura qu'une efficacité très réduite, compte tenu de la vitesse de propagation des fausses informations dont aucune définition satisfaisante, en dépit des efforts de l'Assemblée nationale, n'a pu être trouvée. Plus probablement, face à l'impossibilité de trancher en moins de quarante-huit heures une question mettant en jeu la liberté d'expression, le juge ne prendra pas les mesures de restriction prévues, ce qui reviendra à décerner un brevet de respectabilité à l'information douteuse. À l'opposé, si le juge décide d'appliquer plus sévèrement le référé, il prendra le risque d'interférer dans le débat public en pleine campagne électorale, période durant laquelle la liberté d'expression est par tradition républicaine encore plus respectée. De manière générale, monsieur le ministre, les manipulations d'aujourd'hui sont complexes, multiformes, élaborées comme de vraies stratégies destinées à nuire, et il faut beaucoup de naïveté pour penser qu'un juge de l'urgence sera en mesure de les apprécier dans un délai aussi réduit. Déjà, nous apprenons que les manipulateurs commencent à recourir à de nouveaux subterfuges, destinés aussi bien à contourner les mesures mises en place qu'à s'insinuer toujours plus profondément dans les opinions publiques. Ainsi, les faux comptes sur les réseaux sociaux sont de moins en moins détectables. Des comptes bien réels peuvent même être piratés. Les progrès de l'intelligence artificielle permettent des opérations de manipulation en profondeur directement sur les forums. En un mot, le dispositif proposé, potentiellement dangereux, est probablement déjà dépassé.

En revanche, un effet indirect sur les États se fait sentir, avec une tentation liberticide qui « pourrait être le véritable effet final recherché par les puissances étrangères à l'origine des manipulations de l'information : que d'inciter les gouvernements à prendre des mesures contraires à leurs valeurs démocratiques et libérales ». Monsieur le ministre, comment ne pas mettre en parallèle ces propos et l'article 1 de la proposition de loi, qui suscite une incompréhension si large ? Les autres dispositions du texte, si elles prêtent moins le flanc à la polémique, n'en sont pas moins largement insuffisantes. Les nouveaux pouvoirs confiés au Conseil supérieur de l'audiovisuel par le titre II correspondent à des mesures non expertisées. la capacité de suspendre la diffusion d'une chaîne étrangère fait courir à nos médias le risque de mesures de rétorsion. De telles dispositions auraient plutôt leur place- nous le pensons et nous y travaillerons avec vous, monsieur le ministre -dans le cadre plus vaste de la réforme de l'audiovisuel que le Gouvernement prépare depuis plusieurs mois. La régulation des plateformes constitue bien le sujet central, comme je l'ai dit tout à l'heure. Cependant, la directive e-commerce de 2000 établit un régime d'irresponsabilité des hébergeurs qui prévient toute avancée sérieuse, comme le montre la modestie des mesures prévues dans le texte. Enfin, si le Sénat porte depuis longtemps un grand intérêt à la question de la formation au numérique et aux médias, donc aux dispositions du titre III , il convient de rappeler que des mesures très proches ont été adoptées dès 2011 dans le cadre de l'examen du « troisième paquet télécom », texte dont j'avais l'honneur, déjà à l'époque, d'être la rapporteur. la loi n'a pas vocation à être répétitive ! Aujourd'hui, il manque toujours un plan d'action global et stratégique, comme je l'ai rappelé dans un récent rapport sur la formation à l'heure du numérique,

Aucun des risques que nous avions mis en lumière, notamment sur l'article 1, n'a été pris en compte. En un mot, l'Assemblée nationale a considéré que la position du Sénat était une posture politique, ce que nous regrettons, et n'a pas voulu entendre ce que nous exprimions, à savoir une incompréhension très large- je le répète -de la totalité de nos interlocuteurs, ces nombreuses personnes, tous secteurs confondus, que nous avons auditionnées.

Or, ce modèle imposé, nous n'en voulons pas ! Nous ne voulons pas d'un débat démocratique hystérisé, polarisé, qui déchire les peuples, ce que nous voyons depuis quelques années. Nous voulons- c'est le même sujet -le respect des droits d'auteur. Nous voulons aussi que l'information portée par des rédactions indépendantes puisse vivre.

visant à créer une autorité de déontologie de la presse. La ministre a ainsi indiqué, et l'on ne peut que la suivre, que « le premier rempart contre la désinformation et la manipulation de l'information reste les médias et les journalistes Il s'agit à l'origine d'une proposition de Reporters sans Frontières que son président nous avait exposée lors d'une table ronde au Sénat. Nous suivrons bien sûr avec intérêt cette mission, qui s'annonce bien complexe et ne faisait pas l'unanimité dans la presse. Pour autant, si la solution est une instance de déontologie, il aurait été utile de l'évoquer dès le début de la discussion.

L'expérience allemande n'a pas encore été évaluée, mais elle ne nous paraît pas du tout convaincante, en raison du risque de privatisation de la censure qu'elle fait courir. À ce jour, quelque 87 de mes collègues ont cosigné cette proposition de résolution, et sénateurs issus de tous les groupes du Sénat, ce qui marque bien la nature transpartisane de notre réflexion et le caractère partagé de nos analyses. Ce texte a été adopté à l'unanimité par la commission des affaires européennes sur le rapport d'André Gattolin et de Colette Mélot, En effet, le vrai sujet est bien celui du rôle et du statut des hébergeurs, qui, parfois contre leur volonté, rendent possible la diffusion massive de fausses informations, considérées par des algorithmes aveugles comme autant de sujets susceptibles de susciter l'intérêt, donc une audience monétisée sous la forme de recettes publicitaires. Il faut donc engager dès maintenant des négociations à l'échelon européen, afin de créer un nouveau statut pour ces plateformes et ces moteurs de recherche. Tout cela, vous le voyez, est lié. Les débats en cours en Europe sur les droits d'auteur posent une question très proche. Les oppositions que nous y voyons marquent bien l'importance des intérêts en jeu. Nous ne pouvons pas laisser nos concitoyens, les Français comme les Européens, dépendre d'outils qu'il est si aisé de détourner de leur usage premier. Pour internet, le temps de l'innocence est achevé. Voici venir celui de la responsabilité ! C'est Tim Berners-Lee lui-même, le fondateur du web, qui le dit. Nous avons pleinement conscience que ce chemin n'est pas le plus simple, monsieur le ministre : il est exigeant pour nous tous, beaucoup plus que ne l'est en tout cas l'aventure législative nationale assez fruste qui nous est proposée aujourd'hui. Le Sénat n'a donc aucune raison de modifier sa position de principe. Dans ces conditions, je considère qu'une lecture détaillée

tous les politiques, y compris le Gouvernement et le Président de la République ! Écoutez-moi bien, monsieur le ministre : ceux qui s'attaquent à la presse, comme l'a fait Emmanuel Macron, car il s'est bel et bien attaqué à la presse au moment de l'affaire Benalla,

je pense très sincèrement que, par principe, il ne faut toucher à nos libertés que d'une main tremblante. Les lois qui encadrent notre liberté d'expression ont été écrites patiemment n'ont jamais été des lois de circonstance, sauf dans les pires moments de notre histoire. Et ces lois suffisent largement ! Je suis assez stupéfait du manque de recul historique

Les fausses nouvelles se sont toujours propagées. La grande peur de l'été 1789 n'avait pas besoin d'internet. Une proposition de loi de circonstance ne peut s'inscrire dans la lignée des grandes lois de la III République, celles des années

avec la volonté, non pas de protéger les libertés, mais de beaucoup trop les encadrer. Certes, il faut trouver des solutions pour que les grandes plateformes soient soumises aux lois de la presse, mais ce n'est pas ce que votre proposition de loi prévoit ! Je vous demande donc, monsieur le ministre,

également remarqué que nous avions argumenté sur le fond, très loin des caricatures méchantes qui ont été propagées par la commission des lois de l'Assemblée nationale, auxquelles vous ne souscrivez pas, je l'ai bien compris et vous en remercie. À l'issue de ce débat, j'ai un regret,

Je mets aux voix la motion n° 1, tendant à opposer la question préalable. Je rappelle que l'adoption de cette motion entraînerait

Le scrutin est ouvert.

votre ralliement, certes récent, au soutien de ces deux textes

et que toutes les positions ont pu s'exprimer, la vôtre comme les nôtres. Nous avons mené beaucoup d'auditions, tant à la commission des affaires culturelles qu'à la commission des lois, et tous les interlocuteurs que nous avons

lui mettaient, comme on disait à l'époque, « la pression », Mirabeau lui donna le conseil d'en

en raison du caractère dangereux pour les libertés publiques de la nouvelle procédure de référé anti-, de son caractère inabouti et potentiellement inefficace contre les vraies menaces.

Monsieur le ministre, vous aviez raison : en effet, cette loi sera inefficiente contre les vraies manipulations de l'information, les tentatives clandestines qui altèrent la sincérité des scrutins. Sur ce point aussi, tout le monde est d'accord. Ce n'est pas à travers cette loi que le problème des sera réglé. En revanche, cette loi va créer de nouvelles menaces pour la liberté d'expression et pour la liberté d'informer, ce que nous ne pouvons accepter. Au regard des libertés en jeu, il aurait fallu privilégier l'éducation aux médias, l'appel à la vigilance de chacun face aux contenus diffusés sur internet, plutôt qu'une disposition législative « bricolée » sans grande assurance par l'Assemblée nationale et le Gouvernement, et susceptible de nuire à la diffusion de contenus légitimes. La Commission européenne comme le Conseil de l'Europe invitent à une action politique concertée

monsieur le ministre, que ce n'est pas parce que personne n'a encore légiféré sur le sujet que nous ne devons pas le faire. Les Allemands l'ont fait, mais ils ont pris garde de ne pas toucher au domaine de la loi électorale.

Dans son discours préliminaire sur le projet de code civil, Portalis dit qu'« il faut être sobre de nouveautés en matière de législation, parce que s'il est possible, dans une institution nouvelle, de calculer les avantages que la théorie nous offre, il ne l'est pas de connaître tous les inconvénients que la pratique seule peut découvrir ; qu'il faut laisser le bien, si on est en doute du mieux ; qu'en corrigeant un abus, il faut encore voir les dangers de la correction même ». Pour toutes ces raisons, je vous propose d'adopter cette motion tendant

Je mets aux voix la motion n° 1, tendant à opposer la question préalable. Je rappelle que l'adoption de cette motion entraînerait le rejet de la proposition de loi organique. Je rappelle également que l'avis du Gouvernement est défavorable. En application de l'article 59 du règlement, le scrutin public ordinaire est de droit. Il va y être procédé dans les conditions fixées par l'article 56 du règlement. Le scrutin est ouvert. Personne ne demande

Le scrutin est ouvert.

La séance est reprise. L'ordre du jour appelle la discussion du projet de loi habilitant le Gouvernement à prendre par ordonnances les mesures de préparation au retrait du Royaume-Uni de l'Union européenne (projet n° 9, texte

Madame la présidente, monsieur le président Bizet, monsieur le rapporteur Poniatowski, mesdames, messieurs les sénateurs, un temps suspendus par les échéances internes britanniques et notamment par le vote du budget, les contacts entre négociateurs en vue de la conclusion d'un accord sur le retrait du Royaume-Uni de l'Union européenne ont repris. Comme j'ai déjà eu l'occasion de le dire devant la Haute Assemblée et devant les membres de votre commission spéciale chargée d'examiner ce projet de loi, le temps le temps presse désormais, mais nous continuons à penser qu'un bon accord est possible avec le Royaume-Uni, ce qui serait l'intérêt bien compris des deux parties. De nombreux progrès ont été réalisés depuis le début des négociations avec le Royaume-Uni sur les modalités de son retrait de l'Union européenne, qui doit intervenir le 30 mars 2019. Les négociateurs sont parvenus à se mettre d'accord sur près de 90 % du projet d'accord de retrait, y compris sur des chapitres essentiels de la négociation. Cela concerne en particulier les droits des citoyens européens au Royaume-Uni, qui devraient pouvoir continuer de résider, de travailler et d'étudier au Royaume-Uni dans les mêmes conditions que celles qui sont prévues par le droit européen actuellement. Cela concerne également le règlement financier, puisque le Royaume-Uni accepte de s'acquitter de ses obligations. serait mise en place, qui s'ouvrirait le 30 mars 2019 et s'achèverait le 31 décembre 2020, durant laquelle le Royaume-Uni devrait continuer à appliquer l'intégralité de l'acquis, sans participer au processus décisionnel. Je tiens à cette occasion, une fois encore, à saluer la grande qualité du travail mené par Michel Barnier au nom des Vingt-Sept. Il a permis de maintenir notre unité et d'oeuvrer dans notre intérêt commun. Je sais, à cet égard, que vous vous associez bien volontiers à cet hommage. De fait, c'est bien derrière notre négociateur que nous sommes unis, et non pas contre le Royaume-Uni, comme cela a pu parfois être dit punir celui-ci n'est ni notre intention ni notre intérêt. Vous le savez, rien n'est agréé tant que tout n'est pas agréé. Il reste des difficultés à régler, dont la principale concerne le traitement de la frontière entre les deux parties de l'Irlande. Comme le Royaume-Uni, nous nous sommes engagés à respecter la volonté de tous les Irlandais en évitant de rétablir entre l'Irlande du Nord et la République d'Irlande une frontière dure, qui pourrait menacer la mise en oeuvre des accords du Vendredi saint. Cette question se réglera peut-être dans la relation future entre le Royaume-Uni et l'Union européenne, mais il faut en tout état de cause disposer d'un filet de sécurité, d'une solution de dernier recours, qui consiste en ce que l'Irlande du Nord reste pour l'essentiel dans le marché unique, avec un alignement réglementaire. Cette hypothèse, le Royaume-Uni y a souscrit dès le mois de décembre dernier. Elle implique qu'il puisse y avoir des contrôles, même très allégés, en mer d'Irlande. l'initiative de Londres, les discussions se poursuivent sur la possibilité, pour éviter d'avoir recours à ce filet de sécurité, d'un maintien du Royaume-Uni tout entier dans l'union douanière. Elles sont difficiles, car cela supposerait que celui-ci renonce à passer des accords commerciaux autonomes avec des pays tiers, que nous maintenions le même niveau de concurrence entre les entreprises britanniques et européennes et que nous préservions, par exemple, la possibilité pour les pêcheurs européens de continuer à accéder aux eaux britanniques. Contrairement aux bruits qui se sont multipliés ces derniers jours dans la presse, rien n'est encore acquis. Aussi, même si notre priorité est que l'Union et le Royaume-Uni aboutissent à un bon accord, nul ne peut totalement écarter l'hypothèse d'un échec des négociations, qui serait très coûteux pour l'Union européenne et pour le Royaume-Uni. Il est donc indispensable de nous préparer à tous les scénarios, y compris de façon à pouvoir limiter les conséquences d'un Brexit sans accord, donc sans période de transition. C'est ce que le Conseil européen a demandé aux États membres comme aux institutions, dès le mois de mars dernier. Au niveau de l'Union, une équipe dédiée à ces travaux de préparation a été spécifiquement mise en place au sein du secrétariat général de la Commission. Distincte de l'équipe de Michel Barnier, qui, elle, oeuvre à la conclusion d'un accord, elle identifie les mesures qui devraient être prises en cas de retrait sans accord dans les domaines qui relèvent de la compétence de l'Union. À l'échelon national, il est aussi de notre responsabilité collective, à commencer par celle du Gouvernement, de nous préparer à toutes les hypothèses, y compris celles d'un retrait sans accord, et d'être techniquement prêts si cette hypothèse se vérifiait à la fin de l'année ou, plus tard encore, en cas de refus par la Chambre des communes de ratification d'un accord de retrait. À cette fin, le Premier ministre a demandé à l'ensemble des ministères d'identifier les conséquences d'une absence d'accord et les mesures à prendre, y compris dans le cas où nous aurions très peu de temps pour le faire avant le 30 mars 2019. C'est l'objet du présent projet de loi, présenté le 3 octobre dernier en Conseil des ministres et soumis à l'examen de votre commission spéciale, par lequel le Gouvernement sollicite l'habilitation du Parlement à prendre par ordonnance les mesures nécessaires, soit, pour certaines d'entre elles, en cas d'accord de retrait, soit- et ce sont les mesures les plus nombreuses -en cas d'absence d'accord, dans trois grands blocs de domaines la situation des ressortissants français et, de manière générale, les intérêts français ; la situation des Britanniques en France ; la circulation des personnes et des marchandises. Je souhaiterais en détailler certains aspects.

à prendre en compte certains bénéfices acquis par les ressortissants français durant une période effectuée au Royaume-Uni avant la date de son retrait de l'Union, par exemple pour faire valoir leur période d'activité outre-Manche dans le calcul de leur retraite en France ou continuer à se prévaloir en France de diplômes obtenus au Royaume-Uni. de la question des intérêts français, le projet de loi contient des mesures visant à permettre aux entreprises françaises la poursuite de transferts de produits et matériels de défense à destination du Royaume-Uni, du Royaume-Uni, aux entités françaises d'accéder aux systèmes de règlement interbancaire et de règlement livraison de pays tiers ou de continuer à utiliser des conventions-cadres en matière de services financiers et à sécuriser les contrats existants. Ce sont des domaines techniques, mais j'insiste ici sur une réalité : les entités britanniques n'auront plus accès au passeport financier européen, mais nous voulons que les contrats en cours puissent aller à leur terme et que les entreprises françaises puissent, de leur côté, maintenir leur accès par exemple au marché des changes britanniques. Concernant la situation des Britanniques en France après le retrait, les mesures proposées visent notamment à régir les droits d'entrée et de séjour, l'emploi des ressortissants britanniques exerçant à la date du retrait une activité professionnelle salariée en France, la situation des agents titulaires et stagiaires de la fonction publique française de nationalité britannique, ou encore l'application aux ressortissants britanniques résidant en France au moment du retrait de la législation relative aux droits sociaux et aux prestations sociales. de la circulation des personnes et des marchandises, les mesures proposées doivent permettre d'assurer la continuité du transport par le tunnel sous la Manche ou de pratiquer les contrôles nécessaires à l'entrée de marchandises venant du Royaume-Uni sur notre territoire. À cet égard, certaines mesures seront nécessaires, même en cas d'accord, en vue de la réalisation de travaux de construction ou d'aménagement de locaux, d'installations ou d'infrastructures portuaires, ferroviaires, aéroportuaires et routières qui seront requis d'ici au 31 décembre 2020 par le rétablissement des contrôles de marchandises et des passagers à destination et en provenance du Royaume-Uni. Même si le Gouvernement a pleinement conscience que le recours aux ordonnances est une pratique qui ne recueille pas,, l'assentiment des parlementaires, parlementaires, le choix de l'habilitation, qui permet une plus grande flexibilité, est cependant ici indispensable au regard des enjeux comme de la possibilité de devoir mettre en oeuvre des mesures dans des délais très rapides, à l'approche de l'échéance du 30 mars 2019. Il faudra en particulier que nous puissions ajuster notre dispositif en fonction de l'évolution des négociations, mais aussi des mesures qui seront prises par la Commission pour ce qui relève des compétences communautaires et par les autres États membres. Je tiens tout d'abord à remercier le rapporteur Ladislas Poniatowski et le président Jean Bizet d'avoir relevé cette nécessité et considéré que le Sénat pouvait, au vu du caractère exceptionnel de la situation, accepter l'habilitation sollicitée. Dans ce cadre, le Gouvernement a également pleinement conscience du juste équilibre à trouver entre l'exigence constitutionnelle de précision de l'habilitation prévue par l'article 38 de notre Constitution, d'une part, et le besoin de flexibilité imposée par le contexte des négociations, d'autre part. À cet égard, je renouvelle mes remerciements à votre rapporteur Ladislas Poniatowski de la qualité de son rapport et de sa volonté de préciser le texte. Le dialogue noué avec le rapporteur et votre commission spéciale a permis d'avancer sur la structure même du projet de loi, de façon à mieux faire ressortir la finalité des ordonnances, ou encore sur la reconnaissance de certains diplômes et qualifications professionnelles obtenus après le Brexit. Si la négociation en cours oblige le Gouvernement à garder le champ des options largement ouvert, ouvert, il a entendu la nécessité d'évoquer le maintien en France des ressortissants britanniques ou la poursuite sur notre territoire d'activités économiques liées au Royaume-Uni. Nous aurons ce débat tout à l'heure. Mesdames, messieurs les sénateurs, telles sont les grandes lignes du projet de loi qui vous est soumis aujourd'hui. Le nombre relativement limité de domaines concernés s'explique par la répartition des compétences entre l'Union européenne et les États membres. Plusieurs questions essentielles, comme celles qui sont relatives au transport aérien ou encore à la pêche, seront traitées au niveau communautaire. Je me réjouis que nous puissions maintenant engager le débat en séance publique sur ce texte d'une grande importance pour notre préparation,

sur un texte qui aurait dû être consensuel jusqu'au bout. Vous allez comprendre pourquoi je dis cela. Pour avoir lu en détail tout ce qu'il s'est dit en commission, pu constater que les sénateurs de tous bords se sont montrés particulièrement responsables. Les parlementaires n'aiment pas, en général, les ordonnances. Et pour cause : il s'agit de leur retirer un droit au débat.

Madame la présidente, madame la ministre, mes chers collègues, la presse nationale du mardi 16 octobre 2018 a confirmé que le Gouvernement refusait de rendre public l'avis du Conseil d'État relatif au projet d'ordonnances d'habilitation au sujet du Brexit. C'est exact, car les membres de la commission spéciale du Sénat qui avaient demandé à connaître cet avis ne l'avaient pas obtenu. À l'évidence, le Gouvernement espérait que le Sénat ne serait pas informé des réserves du Conseil d'État au sujet de ce projet de loi. d'un manque de loyauté à l'encontre des parlementaires qui sont appelés à voter sur un texte sans en connaître les tenants et les aboutissants. De plus, c'est contraire à la pratique habituelle, car si effectivement le Gouvernement n'est pas tenu de publier l'avis du Conseil d'État, c'était néanmoins devenu un usage habituel. Quoi qu'il en soit, la presse a eu connaissance de cet avis qui avait été rendu le 27 septembre 2018. Selon le journal, le Conseil d'État regrette que le projet de loi « n'énumère que les têtes de chapitre des domaines pouvant donner lieu à ordonnances, mais sans préciser, dans la plupart des cas, la portée des mesures envisagées. Le Gouvernement explique ces choix par le souci de ménager la position de la France dans les négociations en cours, en préservant ses marges de manoeuvre ». Or, selon le Conseil d'État, la Constitution oblige le Gouvernement à indiquer au Parlement la finalité des mesures envisagées avec une précision suffisante. « Tout en admettant que le projet du Gouvernement s'inscrit dans un contexte très particulier [ ...], le Conseil d'État considère, au stade où il est saisi, que le respect de cette exigence constitutionnelle suppose de préciser davantage l'énoncé de la finalité des mesures ». Dans ces conditions, il apparaît clairement que, selon l'avis du Conseil d'État, ce projet de loi d'inconstitutionnalité. C'est la raison pour laquelle les signataires de la présente motion proposent l'adoption d'une exception d'irrecevabilité.

D'ailleurs, la publication des avis du Conseil d'État était une pratique constante depuis 2015. Toutefois, elle n'est pas obligatoire

ont permis de préciser les finalités des habilitations à légiférer par ordonnance, dans le respect de la jurisprudence du Conseil constitutionnel. Pour ces raisons, la commission spéciale a émis un avis défavorable sur votre motion. Quel est l'avis du Gouvernement ?

pour la seule et unique raison que le projet de loi touche aux relations internationales de la France, à l'instar des projets de loi de ratification d'accords internationaux prévus par l'article 53 de la Constitution, pour lesquels les avis du Conseil d'État ne sont traditionnellement pas rendus publics non plus. Le projet de loi d'habilitation s'inscrit dans un contexte extrêmement particulier et incertain, comme j'ai eu l'occasion de le dire devant vous. Toute la difficulté sur le fond était de concilier la nécessaire précision des ordonnances avec la capacité du Gouvernement à réagir très rapidement en fonction de l'évolution des négociations comme des mesures envisagées par nos partenaires européens et par les Britanniques eux-mêmes en cas d'absence d'accord. L'examen du projet de loi par le Conseil d'État a déjà conduit le Gouvernement à apporter à son texte initial des améliorations, notamment sur les finalités des mesures envisagées. Le Conseil d'État a précisé explicitement dans son avis que, dans la nouvelle rédaction telle qu'elle a été présentée au Sénat, le texte est conforme aux exigences constitutionnelles, eu égard notamment au contexte exceptionnel dans lequel il s'inscrit. C'est pourquoi j'émets un avis défavorable sur cette motion tendant

commission spéciale, hier, des centaines d'Européens résidant au Royaume-Uni et de Britanniques installés dans l'Union ont formé une chaîne humaine devant Downing Street pour demander au gouvernement britannique de garantir leurs droits dans l'hypothèse d'un Brexit sans accord avec l'Union européenne. À l'invitation des organisations The3million et British in Europe, je suis intervenu hier dans l'enceinte du Parlement, à Londres. J'ai souhaité que tout soit entrepris pour sécuriser et préserver les droits des trois millions d'Européens du Royaume-Uni et des deux millions de Britanniques en Europe. C'est également la volonté exprimée par notre gouvernement en de nombreuses occasions. Le cauchemar du Brexit a commencé il y a deux ans, quatre mois et treize jours : 866 jours après le référendum et à J moins 143 de l'échéance, personne ne sait ce que « Brexit » signifie. En tant qu'entrepreneur, on me demande de me préparer ; mais me préparer à quoi ? Le Gouvernement est dans la même situation : il est contraint de nous demander de lui permettre de s'adapter très vite, dès lors que nous saurons ce que le Gouvernement britannique choisira. La raison en est simple : il n'y a pas de consensus au Royaume-Uni sur le projet de sortie. Même si le pire n'est jamais sûr, l'absence d'accord est devenue une option. Personne ne peut plus faire de projets. Pour cinq millions d'Européens, l'angoisse est totale. Il faut que ce cauchemar cesse : il faut donc être flexible et pragmatique, et habiliter le Gouvernement à prendre par ordonnances les mesures de préparation au retrait du Royaume-Uni. Je mets aux voix

Le site internet de l'hebdomadaire résume très bien la duplicité des négociateurs de l'Union européenne dans l'affaire du Brexit. Sous le titre : « Brexit, cette négociation qui n'en est pas une », explique que, malgré une apparente bonne volonté, l'Union européenne ne cherche pas à négocier réellement. En fait, les Européens ont posé d'emblée leurs exigences et ils refusent toute discussion. Ces exigences reposent sur quatre points : premièrement, le refus de traiter séparément la circulation des personnes, des biens, des services et des capitaux le statut des ressortissants européens résidant en Grande-Bretagne ; troisièmement, le solde financier et le paiement par la Grande-Bretagne des projets déjà engagés ; quatrièmement, et enfin, le refus de toute frontière physique entre l'Irlande du Nord et le reste de l'île. Les négociateurs européens savent très bien que cette dernière condition est, à elle seule, un obstacle quasi insurmontable, car, dans le même temps, ils veulent créer une frontière physique avec le reste de la Grande-Bretagne. Cela revient donc à obliger les Britanniques à accepter un dépeçage de leur pays, lequel serait littéralement coupé en deux par une véritable frontière. résume très bien la finalité des responsables : ils veulent absolument que les Britanniques perdent tous leurs avantages et qu'ils vivent moins bien, tout cela afin qu'ils regrettent leur départ. À la veille des élections européennes, leur seul but est de faire croire à nos concitoyens que l'évolution vers une Europe fédérale serait la seule solution de bon sens pour l'avenir. Ainsi, l'impasse actuelle des négociations sur le Brexit est en très grande partie due à la stratégie politicienne des dirigeants de l'Union européenne. Le président Macron est à la pointe de la coalition, qui essaie de saboter le Brexit en « pourrissant » les négociations. Le Gouvernement français ferait vraiment mieux de chercher honnêtement des solutions plutôt que de mettre de l'huile sur le feu par son intransigeance. Cela justifie donc l'adoption d'une motion tendant à opposer la question préalable, conformément à l'article 44, alinéa 3, du règlement du Sénat. Y a-t-il un orateur contre ?

représentent 3 % du PIB français ; en outre, chaque année, quelque 32 millions de personnes et 4,2 millions de poids lourds franchissent la Manche soit par le tunnel, soit en bateau, soit en avion ; enfin, 4 millions de Britanniques se rendent chaque année sur le territoire français.

Quel est l'avis du Gouvernement ? Notre objectif est, aujourd'hui comme hier, de parvenir au meilleur accord possible pour le Royaume-Uni et pour l'Union européenne. Le projet de loi présenté en conseil des ministres ne constitue pas un acte de défiance, ni à l'encontre du Royaume-Uni ni à l'encontre des négociations : celles-ci se poursuivent et le négociateur de l'Union a l'entier soutien du gouvernement français. Toutefois, l'hypothèse d'un échec des négociations, ou celle d'une absence de ratification par l'une des deux parties, ne peut être exclue. C'est la raison pour laquelle la France, tout comme les vingt-six autres États membres et les institutions de l'Union européenne, mais aussi le Royaume-Uni, pour ce qui le concerne, se prépare à toutes les éventualités, y compris une absence d'accord. est le sens du projet présenté au conseil des ministres, qui vise à permettre au Gouvernement de prendre, par ordonnances, les mesures nécessaires, soit, pour certaines d'entre elles, en cas d'accord de retrait, soit en cas d'absence d'accord. Contrairement à ce que vous laissez entendre, madame Kauffmann, nous n'essayons ni de « saboter le Brexit » ni de « pourrir les négociations » ; nous veillons simplement à préserver les intérêts de notre pays, quelles que soient les hypothèses. C'est la raison pour laquelle le Gouvernement émet un avis défavorable à la motion tendant à opposer la question préalable. vote. Madame la présidente, dès l'annonce du résultat du référendum en 2016, j'ai pris avantage de mes différents déplacements dans de nombreux pays de l'Union européenne pour interroger les gouvernements et les parlementaires et savoir s'ils pouvaient être favorables à la restriction de la liberté de circulation au sein de l'Union européenne, comme le souhaitaient les Brexiters. Leurs réponses ont été unanimement contre la moindre restriction à cette liberté au sein de l'Union européenne, qui est une liberté fondamentale. J'ai également observé une unanimité, à la fois pour défendre le statut des trois millions d'Européens vivant au Royaume-Uni, Royaume-Uni, et pour que les Britanniques assurent leurs engagements financiers pris en qualité de membre à part entière de l'Union européenne. Enfin, j'ai constaté la même l'unanimité pour que les accords du Vendredi saint soient préservés. En effet, l'Union européenne a permis que le conflit en Irlande du Nord prenne fin. Elle a investi des milliards d'euros pour soutenir le développement de l'Irlande du Nord. La visite du groupe de suivi sur le Brexit, présidée par Jean Bizet, à Belfast, nous a permis d'observer que la situation restait tendue. Il faut donc éviter toute frontière physique entre l'Irlande du Nord et la République d'Irlande ; sinon, la menace d'un retour au conflit ne peut être exclue. Les négociations conduites par Michel Barnier pour l'Union européenne sont exemplaires. La position de l'Union européenne n'a jamais varié. En réponse aux orateurs qui cherchent à accabler Emmanuel Macron, adoptant les mots des « ultra-Brexiters », je rappelle que celui-ci n'était pas Président de la République lorsque cette position de l'Union européenne a été adoptée. L'Union européenne a été fidèle à sa devise : « Unie dans la diversité Durant la campagne, les Brexiters annonçaient que, sitôt le Brexit voté, l'Union européenne imploserait. Aujourd'hui, c'est plutôt le contraire qui pourrait bien se passer. Je ne comprends pas que des parlementaires français puissent reprendre les arguments des Brexiters les plus agressifs : eux ne se soucient ni de l'intérêt de la France, ni de celui de l'Union européenne. Voilà pourquoi nous devons faire bloc avec le Gouvernement et voter contre cette motion.

le Gouvernement s'intéresse au sort des Britanniques installés en France : or nous savons que, si nous ne traitons pas cette question positivement, si nous ne leur garantissons pas le droit au séjour ou leurs acquis sociaux, leurs acquis sociaux, il n'y aura pas de réciprocité pour nos concitoyens installés en Grande-Bretagne. C'est l'une des raisons, parmi beaucoup d'autres, qui nous incite à ne pas voter cette question préalable.

Madame la présidente, madame la ministre, mes chers collègues, en 2016, les Britanniques choisissaient de délier leur destin de celui de l'Union européenne. En votant en faveur du, ils ont choisi le « grand large », selon la fameuse expression churchillienne. Le choc fut rude même si nous savions les limites d'une adhésion en demi-teinte le Royaume-Uni avait renégocié sa contribution financière, s'était exclu de Schengen, de l'euro ou encore de la Charte des droits fondamentaux. Pendant plus de quarante ans de vie commune, l'Angleterre a toujours eu un pied dehors, un pied dedans. Aussi, il n'est pas surprenant que cette dichotomie ressurgisse à propos de l'accord de retrait, jusqu'à rendre- peut-être -celui-ci impossible pour des considérations qui ne sont même plus d'ordre technique. C'est bien dommage

avons tous bien compris que Theresa May essayait de naviguer entre les europhobes de son propre parti et ceux qui regrettent le Brexit, tout cela avec, en point d'orgue, la question de la frontière entre la République d'Irlande et l'Irlande du Nord. Et pour ne rien arranger, les nationalistes écossais ne sont pas en reste lorsqu'ils soutiennent l'idée d'un nouveau référendum. Comme l'a très justement souligné le Président de la République à l'issue du dernier Conseil européen : « Ce Ce n'est pas à l'Union européenne de faire des concessions pour trouver des solutions à un problème politique interne britannique. » Le groupe du RDSE partage cette position. Il revient au Royaume-Uni d'assumer ses difficultés intérieures et de ne pas demander l'impossible pour tenter de les résoudre, comme ce fut le cas avec le plan de Chequers, une sorte de marché unique à la carte. Bien sûr, il ne s'agit pas pour autant de méconnaître la très délicate question irlandaise, bien au contraire. La construction européenne a dans ses gênes l'idée de paix. Le format du retrait britannique ne doit en aucun cas menacer les accords du Vendredi saint, tout le monde en convient. C'est pourquoi l'idée du prôné par Michel Barnier, le filet de sécurité entre l'Irlande du Nord et l'Union européenne, est une très bonne option. Espérons seulement qu'elle gagne rapidement du terrain outre-Manche. J'en profite pour saluer le travail remarquable de notre compatriote négociateur en chef de la Commission, qui ne ménage pas sa peine pour trouver le meilleur compromis et qui s'emploie à présenter le visage d'une Europe à vingt-sept Quoi qu'il advienne, avec ou sans accord, le retrait étant irréversible, l'Union européenne, et au sein de celle-ci notre pays, doit s'y préparer. Le Conseil européen l'a rappelé depuis 2017 lors de chacune de ses réunions. Nous y sommes aujourd'hui. La mise en oeuvre de l'article 50 du traité sur l'Union européenne étant une première, ses conséquences soulèvent des inquiétudes, s'agissant en particulier de la libre circulation des personnes et des marchandises. Demain, le Royaume-Uni sera un État tiers. Les enjeux sont nombreux pour les citoyens, les expatriés, les couples mixtes, dont la circulation et les droits pourraient être un temps entravés. Quant aux marchandises, on imagine aisément, en cas d'impréparation, les difficultés que pourrait avoir le rétablissement des frontières lorsque l'on sait, par exemple- je tiens à le redire que chaque année transitent 25 millions de tonnes de marchandises par le tunnel sous la Manche. Le projet de loi d'habilitation qui nous est soumis cet après-midi doit anticiper ces situations. Compte tenu du contexte que nous avons tous évoqué, évoqué, celui de négociations non abouties- tout au moins dans les délais fixés initialement -, le projet de loi présente la particularité de proposer des habilitations contenant des mesures de portée très générale, voire peu précises quant à leurs finalités. Le Conseil d'État s'en est d'ailleurs ému, mais il faut reconnaître, madame la ministre, que l'équation est complexe. On mesure bien les contraintes qui entourent ce texte : des négociations en suspens- je viens de le rappeler -qui commandent une certaine flexibilité au sein de ces ordonnances, la nécessité également de tenir compte des dispositions qui seront prises par le Royaume-Uni, par l'Union européenne et par chacun des États membres. Pour toutes ces raisons, le groupe du RDSE estime que ces ordonnances se justifient, même si, en tant que parlementaires, nous n'en sommes pas très friands, car, disons-le, elles comportent souvent une part d'inconnue. La commission spéciale a en tout cas entrepris un travail de clarification et de consolidation des quatre articles du projet de loi, qui va, pour l'essentiel, dans le bon sens. Je pense en particulier aux amendements à l'article 3 concernant le régime applicable aux travaux de construction et d'aménagement qui seront rendus nécessaires par le rétablissement de contrôles aux frontières. Cet article concerne près d'une dizaine de codes et des mesures allant du permis de construire au travail de nuit, en passant par les obligations environnementales. Si l'urgence peut conduire à contourner provisoirement le droit commun, l'allégement des procédures doit néanmoins être borné par le respect des droits et des libertés garantis par la Constitution. C'est un apport très utile de la commission spéciale que je souhaitais souligner. Je regrette donc l'amendement du Gouvernement tendant à introduire le mot « notamment ». Je pensais naïvement que ce mot était à proscrire dans un texte de loi, mais peut-être est-ce pour nous signaler que la liste des adaptations ou des dérogations, déjà longue, est incomplète. Nous en débattrons, madame la ministre, lors de la discussion des amendements. Mes chers collègues, dans cette épreuve qui secoue l'Europe, les États membres ont leur part de travail à fournir pour protéger nos concitoyens et nos intérêts. Le groupe du RDSE, profondément attaché au projet européen, sera au rendez-vous des mesures qui faciliteront la concrétisation d'une Europe à Et, au-delà, nous espérons qu'un divorce à l'amiable est encore possible, afin de réussir au mieux la prochaine étape, le cadre des relations futures entre l'Union européenne et le Royaume-Uni. La parole

Kern. Madame la présidente, madame la ministre, monsieur le président de la commission spéciale, mesdames, messieurs les rapporteurs, mes chers collègues,

Dans moins de cinq mois maintenant, le Royaume-Uni ne sera plus membre de l'Union européenne. C'est une réalité à laquelle nous avons encore, parfois, du mal à faire face, et le groupe Union Centriste, que j'ai l'honneur de représenter, particulièrement attaché à la construction européenne, ne s'y résout pas de gaîté de coeur. Il faut bien, malgré tout, s'y résoudre, et tâcher de prendre des mesures qui préservent au mieux les intérêts de notre pays et de l'Union. L'objet du projet de loi que nous examinons aujourd'hui est de permettre au Gouvernement de prendre, par ordonnances, des dispositions tant structurelles que d'urgence visant à adapter notre pays aux conséquences du retrait britannique., le Parlement n'est évidemment pas favorable, ou alors très rarement, au recours aux ordonnances. Or il est ici de l'impérieuse nécessité que certains aspects essentiels soient anticipés, et les délais impartis nous paraissent justifier cette procédure. Parmi les multiples conséquences du Brexit se pose la question de l'avenir du « passeport européen » pour les établissements financiers. Après le retrait du Royaume-Uni, les établissements financiers britanniques vont en effet perdre leur « passeport financier européen Il ne leur sera donc plus possible de bénéficier de la procédure de « passeportage » concernant les prestations de service, qui prendront fin. Dans ce contexte, le Royaume-Uni élabore actuellement un projet de régime temporaire, qui pourrait permettre à certaines entités bénéficient du passeport européen de se prévaloir, pour certaines activités, d'un régime ne nécessitant pas d'agrément nouveau. Pour l'instant, il n'existe toutefois pas de proposition similaire pour l'Union européenne, qui attend le résultat des négociations pour statuer, même si d'autres possibilités pourraient être envisagées, au regard des textes existants, pour que le Royaume-Uni puisse exercer dans l'Union européenne. Tout dépendra bien évidemment du résultat des négociations en cours. Cela impose, pour les contrats en cours, un transfert vers des entités relevant du droit européen, avec les incertitudes liées à une mise en oeuvre pratique, surtout quand on connaît les subtilités juridiques françaises concernant les notions de novations et de cession de contrat. L'incontournable réalité pratique est que le temps court et qu'il convient se préparer au pire des scénarios l'impossibilité de poursuivre les relations financières existantes. Au-delà de la problématique financière, j'insiste sur le fait que le Brexit risque d'entraîner une forte désorganisation économique, dont les conséquences seront notamment visibles dans la région du Grand Est et, partant, dans la collectivité d'Alsace. La sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne aura en effet un très fort impact sur les entreprises de la région, alors même qu'elles ont exporté outre-Manche pour près de 5 milliards d'euros de marchandises, soit 13,6 % du total des exportations. Si les gros opérateurs de commerce ont pris les devants, cette situation reste problématique et fastidieuse pour les PME, notamment dans les domaines agroalimentaire et viticole. ne sont pas forcément rompues aux règles de l'Organisation mondiale du commerce, l'OMC, qui s'appliqueraient au cas où le Royaume-Uni deviendrait un pays tiers, sans autre cadre juridique préalablement négocié. du groupe Union Centriste restent très attentifs à l'évolution des négociations en cours entre Londres et Bruxelles. Si nous gardons espoir quant à la conclusion d'un accord, nous souhaitons que toutes les mesures nécessaires soient prises pour faire face à ces diverses éventualités. C'est pourquoi nous voterons ce texte, en demeurant vigilants quant à la mise en oeuvre des ordonnances qu'il prévoit, dans le respect des compétences du Gouvernement et du Parlement. Très bien

Quoi qu'il arrive, le Royaume-Uni ne sera plus un État membre de l'Union européenne le 30 mars 2019, c'est-à-dire demain. Bien que l'actualité récente nous apporte un peu d'espoir, avec la perspective d'un accord sur la frontière irlandaise, nous ne devons pas nous voiler la face

que je souhaite souligner ici, un Brexit sans accord marquerait la victoire de la division et de l'entêtement entre deux amis, entre deux partenaires. Nous ne pouvons concevoir cette issue, tant il nous semble que l'avenir du Royaume-Uni est lié de façon inaltérable à l'Union européenne. Nous ne pouvons imaginer qu'un ancien membre de l'Union, un pivot historique du concert européen, un allié essentiel de la France soit traité comme n'importe quel État tiers ce n'est pas dans l'intérêt du Royaume-Uni, ce n'est pas dans l'intérêt de l'Union européenne, ce n'est pas dans l'intérêt de la France. N'oublions pas que nous sommes en train de perdre la deuxième économie d'Europe, alors que nous sommes confrontés à une situation mondiale des plus dangereuses. Un Brexit sans accord est également une menace majeure pour les intérêts de nos compatriotes expatriés. La communauté française est nombreuse au Royaume-Uni plus de 300 000 personnes, parmi lesquelles nombre d'étudiants et de jeunes travailleurs. Ce projet de loi a pour objet de préserver leurs intérêts, en traitant de leurs droits sociaux et de la reconnaissance des qualifications entre nos deux pays. Comment imaginer qu'un étudiant français Erasmus ou, demain, un jeune Français étudiant à Oxford puisse se voir refuser son diplôme en France ? À cet égard, je salue l'action de notre commission spéciale, qui a prévu d'inclure dans l'habilitation les diplômes et qualifications professionnelles complémentaires, même si les formations débutent après le retrait du Royaume-Uni de l'Union européenne. Exact ! Enfin, un Brexit dur est une menace pour nos intérêts économiques et sécuritaires. Le Royaume-Uni fait partie de nos dix principaux partenaires commerciaux, et il est l'un des rares pays développés avec qui nous ayons encore un excédent commercial. La place financière de Londres est toujours un acteur incontournable dans le financement de l'Union européenne et de la zone euro. Nous devons préserver une relation économique étroite et réciproque entre nos deux pays, dans tous les domaines. Pour ce qui concerne les échanges financiers, il faudra trouver un régime satisfaisant pour remplacer le fameux passeport financier. Il faudra également trouver des solutions viables pour nos pêcheurs du nord, dont l'activité dépend, pour une bonne part, des eaux britanniques. De plus, il faudra trouver une réponse pérenne à la question des échanges le tunnel sous la Manche. Ce projet de loi d'habilitation nous permettra de répondre à ces questions dans l'urgence d'un. Mais la France devra oeuvrer avec ses partenaires européens pour trouver des solutions communes et pérennes.

Le Royaume-Uni est et restera un partenaire indispensable de la France et de l'Europe en matière de défense et d'armement. Cette coopération politique étroite ne doit pas achopper sur des détails techniques. - République et Territoire espèrent que le Gouvernement n'aura pas à prendre les ordonnances dont nous débattons. Elles signifieraient l'échec du compromis et de la négociation. Elles signifieraient la mise en oeuvre d'un régime d'expédients et de rustines, en lieu et place d'un accord solide et pérenne. Elles signifieraient enfin une cassure irrémédiable, que nous ne souhaitons pas, avec le Royaume-Uni, un grand pays, partenaire historique de la France et de l'Europe. de l'Europe. Nous voterons bien entendu en faveur de ce texte, sous réserve des conclusions de la discussion qui va suivre. La commission spéciale a travaillé de manière consensuelle.

Notre priorité doit demeurer la préservation des intérêts des citoyens européens et de nos entreprises européennes. Veillons à ne pas brader l'intégrité du marché unique, la libre circulation des personnes,

Il est urgent de prendre les dispositions nécessaires pour tirer les conséquences d'une sortie, avec ou sans accord, ratifiée ou non par le Parlement britannique et le Parlement européen. Nous devons donc être pragmatiques : d'où le choix des ordonnances, que nous soutenons.

Madame la présidente, madame la ministre, mes chers collègues, le 30 mars 2019, le Royaume-Uni quittera l'Union européenne et deviendra donc un pays tiers. quel que soit le scénario envisagé, ce changement aura des impacts importants pour les entreprises, les administrations et les citoyens européens et britanniques. En effet, comme le souligne le rapport, les exportations vers le Royaume-Uni représentent 3 % de notre PIB. Environ 30 000 entreprises françaises exportent des marchandises ou des services vers la Grande-Bretagne, et 4 millions de Britanniques se rendent chaque année sur notre territoire. Au-delà des questions techniques et juridiques qu'il soulève, le Brexit est une première dans l'histoire européenne. Et comme l'a très bien identifié le groupe de suivi du Sénat, l'Union européenne doit aujourd'hui gérer une procédure de retrait en deux étapes, qu'elle n'a ni choisie ni décidée. Séisme politique et juridique, le Brexit interroge le concept même d'une « union sans cesse plus étroite » entre les peuples de l'Europe

que la marche en avant du projet européen soit pour autant remise en question ou revisitée. C'est dans ce contexte que nous pouvons aborder le retrait du Royaume-Uni, puissance politique, économique et militaire de premier plan, qui jouissait déjà d'un statut extrêmement dérogatoire par rapport aux autres États membres.

du rapport regrettent une préparation tardive « des administrations et de la mise en adéquation des moyens budgétaires [qui] doivent aller de pair avec des actions de sensibilisation des acteurs intéressés aux conséquences du Brexit En effet, alors que les problématiques sont énormes et diverses, il semble que l'Union européenne et les États membres ont préféré jouer la carte d'une remise en cause du Brexit, plutôt que celle de la négociation d'une sortie ordonnée du Royaume-Uni.

peu instrumentalisé l'Ulster, afin de faire pression sur les négociations, ne peut être balayée d'un revers de la main. Or cette question irlandaise est essentielle, historiquement, politiquement et économiquement. Le retour à une frontière physique « dure » est impossible. Les Irlandais ne reviendront pas sur les accords du Vendredi saint, qui, en 1998, ont mis fin à des décennies de conflits et de violences. Pour eux, il n'y aura pas d'accord de retrait sans quant aux relations entre l'Ulster et la République d'Irlande, aujourd'hui normalisées. L'idée d'une frontière au milieu de la mer d'Irlande, pour maintenir artificiellement l'Ulster dans la zone Europe, est tout à fait inacceptable pour la Grande-Bretagne et l'Irlande, toute forme d'annexion

l'Union européenne ne doit pas spéculer sur les dissensions internes au Royaume-Uni. Où en sommes-nous aujourd'hui ? Alors que, la semaine dernière, les négociations semblaient être dans l'impasse, que l'hypothèse d'un Brexit sans accord était de plus en plus plausible, le secrétaire d'État britannique chargé du Brexit a estimé, dans une lettre adressée aux parlementaires, qu'un accord sur la sortie de l'Union européenne pouvait être scellé d'ici au 21 novembre prochain. Il a même affirmé que l'accord de retrait était désormais réglé Comme l'a souligné le Conseil européen de juillet 2018, un retrait du Royaume-Uni sans accord nécessiterait l'adoption, par l'Union comme par les États membres, dans leur champ de compétences, de mesures de contingence. C'est dans ce contexte mouvant et incertain que nous sommes appelés aujourd'hui à nous prononcer sur la demande d'habilitation formulée par le Gouvernement en vue de combler le vide juridique que provoquerait un Brexit sans accord. Ce projet de loi d'habilitation, au champ d'application extrêmement large et au contenu particulièrement flou- plusieurs orateurs l'ont rappelé, comme l'avait souligné le Conseil d'État dans son avis -, a pour objet la situation des Français installés au Royaume-Uni et des Britanniques installés chez nous, la gestion des flux de personnes et de marchandises et l'aménagement, en urgence, des lignes ferroviaires, des ports et des aéroports français. Nous approuvons les conclusions de M. le rapporteur. La législation par voie d'ordonnances n'est pas une bonne méthode, et, dans ce cas précis, le Gouvernement demande quasiment un blanc-seing au Parlement.

nous comprenons l'exigence de flexibilité qu'exprime le Gouvernement face à une situation exceptionnelle, mais les sénateurs du groupe CRCE resteront extrêmement vigilants, en particulier au sujet des mesures prises sur le fondement de l'article 3,

La Grande-Bretagne est un allié historique. C'est aussi l'un de nos principaux partenaires économiques. Ces chiffres ont été rappelés : 30 000 entreprises françaises y exportent l'équivalent de 3 % de notre PIB. Il s'agit d'une histoire humaine : près de 200 000 Britanniques vivent en France, et plus de 300 000 Français se sont installés chez notre voisin. Le 23 juin 2016, nos amis britanniques ont décidé de quitter l'Union européenne. On peut le regretter, mais nous devons respecter ce choix souverain, que le gouvernement de Mme May a légitimement traduit en activant l'article 50 du traité sur l'Union européenne. En conséquence, le 30 mars 2019, sauf si les vingt-sept États membres décident, à l'unanimité, de fixer une date ultérieure, ce qui paraît fort peu probable, la Grande-Bretagne deviendra un pays tiers. En l'état, la plus grande incertitude demeure quant à un accord de retrait négocié, d'autant qu'il devra être approuvé tant par le Parlement européen que par le Parlement britannique, au sein duquel la Première ministre peine à trouver une majorité, quelle que soit l'option qu'elle proposerait. proposerait. Bien sûr, nous saluons l'action de Michel Barnier, qui conduit avec diplomatie et fermeté les discussions au nom de l'Union européenne. À ce jour, les négociateurs disent s'être mis d'accord sur 90 % à 95 % des sujets. Reste cependant un point de blocage : la frontière irlandaise. De nouvelles propositions ont été faites à la Grande-Bretagne pour dépasser cette difficulté.

des ressortissants britanniques et français à cheval sur les deux pays, qui se trouvent dans une situation juridique incertaine et qui voient leurs droits à circuler, séjourner et travailler remis en cause. Ce sont aussi des entreprises dont les exportations sont entravées, des embouteillages monstres à l'entrée du tunnel sous la Manche, notamment pour le 1,6 million de Ce sont des contraintes techniques considérables pour les ports qui voient transiter 3,6 millions de camions par an. C'est la restauration des droits de douane et des contrôles phytosanitaires. C'est la délivrance de visas pour les 4 millions de Britanniques qui viennent en France chaque année. Bref, c'est le chaos Face à ces nombreuses menaces, face au risque qu'il n'y ait pas de période de transition, nous ne pouvons que souscrire à la demande d'habilitation émise par le Gouvernement. Il s'agit de préparer cette échéance par voie d'ordonnances, pour en atténuer les effets, dissiper les craintes des personnes concernées et fluidifier nos échanges Des mesures urgentes et temporaires doivent bel et bien être adoptées. Madame la ministre, vous le savez, le Parlement n'apprécie guère les ordonnances, et il y en a déjà eu beaucoup depuis le début de ce quinquennat. De plus, en refusant de publier l'avis du Conseil d'État, vous avez alarmé les sénatrices et sénateurs membres de la commission spéciale. Y aurait-il quelque chose à cacher ? Nous entendons vos arguments

ce que le Conseil d'État traduit, en termes plus policés, en soulignant que le périmètre du projet de loi est trop large et que la portée des mesures reste imprécise.

Que le Brexit soit ou, il sera douloureux, y compris pour la France. Plusieurs questions majeures vont se poser pour nos concitoyens. Imagine-t-on une politique des visas entre la France et le Royaume-Uni ?

Il est important de garantir une continuité des droits pour nos concitoyens, tout comme pour les sujets de Sa Majesté. Aussi le Gouvernement doit-il s'assurer, par ces ordonnances, des principes de réciprocité et de proportionnalité, ainsi que du respect des droits fondamentaux et des libertés constitutionnelles.

automobile, pour avoir rencontré, récemment, le patron d'une PME de ce secteur. La Grande-Bretagne exporte chaque année un million de véhicules dont les pièces détachées viennent en grande partie du continent.

Nos collectivités territoriales, quant à elles, ne peuvent être laissées seules en première ligne face aux acteurs économiques de leurs territoires. Les régions, départements et agglomérations concernés agiront, mais le Gouvernement devra dire rapidement de quelle manière il les accompagnera.

accueillir de nouveaux douaniers et des agents des services vétérinaires et phytosanitaires, dont le nombre, soit dit en passant, est insuffisant. Le rétablissement d'une frontière sur les ports de la Manche va coûter cher. Dans ce domaine également, il faut donc que le Gouvernement précise rapidement de quelle manière il contribuera au financement des travaux indispensables et quels moyens humains il mettra à leur disposition.

C'est une véritable inquiétude pour leur attractivité et leur capacité à mobiliser des fonds européens, que nos amis belges et néerlandais ont déjà largement consommés. C'est un non-sens quand on regarde une carte du nord de l'Europe, attestant que les ports français sont plus proches de l'Irlande.

Aussi attendons-nous du Gouvernement qu'il obtienne de la Commission le rattachement de nos ports de la Manche à ce corridor mer du Nord-Méditerranée. Ce projet de loi n'est qu'une étape sur la route qui sépare la Grande-Bretagne et l'Union européenne.

Le Brexit représente un défi majeur. La France a une responsabilité particulière pour défendre le marché unique et les valeurs de l'Union européenne. Il y va des droits de nos concitoyens, de la force de nos entreprises, de l'attractivité de nos territoires et de notre image diplomatique.

Madame la présidente, madame la ministre, monsieur le président de la commission spéciale, monsieur le rapporteur, mes chers collègues, le 23 juin 2016, le peuple britannique a fait le choix de quitter l'Union européenne. S'il ne nous appartient évidemment pas de remettre en question cette décision souveraine, permettez-moi de rappeler de nouveau à quel point nous la regretterons profondément. Avec le départ de l'un de ses membres les plus éminents, c'est une part de l'âme et du génie de notre continent, comme de sa force collective, qui se dissocie de notre édifice commun. Le Brexit, par sa radicalité, interpelle tous ceux qui sont sincèrement attachés à la construction européenne. Il oblige, si l'on veut mener à bien son indispensable refondation, à exercer un devoir d'inventaire lucide sur l'Europe que nous avons bâtie depuis soixante ans. Au-delà des réflexions qu'il a suscitées sur l'avenir de l'Union, le Brexit doit également nous conduire à des considérations plus prosaïques. En effet, nous sommes aujourd'hui dans une situation inédite. Après avoir cherché à organiser la convergence entre ses États membres pendant plusieurs décennies, l'Union européenne doit désormais trouver la voie appropriée pour gérer la divergence à venir entre le Royaume-Uni et le continent. Après quarante ans d'imbrication de plus en plus poussée de nos systèmes économiques respectifs dans le cadre du marché unique, de l'union douanière et de nos diverses politiques communes, nul ne peut en effet ignorer que ce processus emportera des conséquences négatives des deux côtés de la Manche et de la mer du Nord

S'agissant des marchandises, la remise en place de contrôles douaniers, notamment phytosanitaires et vétérinaires, perturbera immanquablement les chaînes d'approvisionnement et de production dans de très nombreux secteurs. La France, en raison de sa géographie et de ses liens économiques étroits avec le Royaume-Uni, comptera au nombre des États membres les plus touchés. Un simple coup d'oeil au volume impressionnant du trafic transitant par le tunnel sous la Manche, qui représente un quart de la totalité des échanges entre le Royaume-Uni et les Vingt-Sept, permet d'en prendre la mesure. L'activité de nos ports, particulièrement en Bretagne, en Normandie et bien sûr dans les Hauts-de-France, ma région, subira également de plein fouet l'impact du Brexit.

car elle accentue encore le risque, déjà existant, de déport des activités vers les ports belges et néerlandais, où les autorités semblent, selon les professionnels que nous avons auditionnés, plus souples, plus réactives et plus avancées aujourd'hui que la France dans la préparation conjointe du Brexit avec le secteur privé. Les conséquences économiques et sociales seront réelles, quel que soit le dénouement des discussions en cours, mais elles seront encore amplifiées en cas de, un scénario qui ne peut plus être écarté, au vu de au vu de la situation politique intérieure au Royaume-Uni, ainsi que de l'échec du sommet de Salzbourg et du dernier Conseil européen. À cinq mois de la sortie effective du Royaume-Uni, le brouillard qui entoure l'issue des négociations concernant l'accord de retrait n'est pas levé levé et empêche toujours d'entrevoir les contours de nos relations futures avec Londres. En conséquence, il apparaît indispensable d'anticiper le pire et de se préparer à un retrait sans accord, afin d'en minimiser autant que possible l'impact. est l'objet du projet de loi qui nous est soumis par le Gouvernement, qui doit permettre de faire face, dans les domaines qui relèvent de la compétence nationale, aux conséquences du Brexit, que celui-ci soit négocié

en précisant ses finalités, tout en lui conservant la flexibilité nécessaire pour réagir aux événements. Comme parlementaire, j'ai, en revanche,

Celle-ci dépendra avant tout des moyens concrets que le Gouvernement lui allouera et de la rapidité d'action de l'État, pour apporter une réponse appropriée aux problèmes d'ores et déjà identifiés sur le terrain. Tout retard pris aujourd'hui sera en effet très difficile à combler d'ici au 29 mars 2019, date à laquelle nous devons être prêts en cas de. L'urgence est réelle. Elle concerne les nombreux investissements et les procédures nécessaires à la mise en place de contrôles douaniers efficaces et aux ressources humaines qui devront être mobilisées en conséquence.

stade. Il doit également être présent pour accompagner nos territoires, particulièrement ceux du littoral atlantique, et nos entreprises, notamment les PME, face aux turbulences qu'ils auront à traverser. D'autres États membres ont d'ores et déjà engagé cette démarche ; la France doit le faire sans plus attendre et amorcer une véritable logique de partenariat avec les acteurs de terrain, au niveau tant administratif que technique.

Madame la présidente, madame la ministre, monsieur le président de la commission spéciale, monsieur le rapporteur, mes chers collègues, le 23 juin 2016, le Royaume-Uni a donc choisi de sortir de l'Union européenne. Il redeviendra un pays tiers le 30 mars prochain à minuit,

Dans cette hypothèse, la plus négative pour toutes les parties, il n'y aura donc pas de période de transition. Pour tenter de se préparer, de préserver les acquis des Français et des Britanniques, d'assurer une continuité en matière de libre circulation des biens et des personnes dans les meilleures conditions possible et sous réserve de réciprocité, le Gouvernement nous propose aujourd'hui de l'autoriser à légiférer par ordonnances. Dans le contexte d'urgence que nous connaissons, le groupe Union Centriste apportera son soutien à ce projet de loi, qui bien sûr prendra en compte les amendements de notre commission spéciale.

et nos exportations sont d'ores et déjà affectées par une demande intérieure britannique en baisse, à cause de la chute de la livre sterling et de l'augmentation du coût du pétrole. Les secteurs les plus pénalisés dans les mois et les années à venir devraient être l'automobile, avec un manque à gagner estimé à plus de 1 milliard d'euros, les outils et l'équipement, l'agroalimentaire ou la pharmacie. On peut penser que les plus grandes entreprises disposeront de l'ingénierie nécessaire pour faire face aux difficultés que cette situation ne manquera pas de provoquer, mais qu'en sera-t-il de nos PME ?

notamment pour développer les compétences nécessaires et gérer les ruptures d'approvisionnement, ainsi que les certifications. Chacun est bien conscient que les accords ultérieurs de libre-échange avec l'Union européenne seront déterminants, mais ils ne seront conclus que dans plusieurs années. Le gouvernement britannique est allé jusqu'à prévoir une bonne dizaine d'années pour mener à bien les diverses négociations déclenchées par le Brexit, même dans un scénario optimiste, qui verrait le Royaume-Uni discuter avec l'Union européenne d'un accord de libre-échange similaire à celui liant le Canada au bloc européen. S'ouvre donc pour nous tous, Européens, une longue période d'incertitude, dont les conséquences seront lourdes pour les nombreuses entreprises françaises qui commercent avec le Royaume-Uni, mais aussi pour les produits britanniques, qui entreront désormais dans une nouvelle Union européenne.

Alors que l'Union européenne est déstabilisée et remise en cause dans sa gouvernance comme dans ses modes de fonctionnement, en raison de ce qu'il faut bien appeler ses non-choix, les signes d'éclatement que traduisent le Brexit et la montée des populismes fragilisent encore le projet de reconstruction de la République, qui est aujourd'hui bien isolé. Votre tâche sera lourde, madame la ministre, mais les membres du groupe Union Centriste seront à vos côtés. Nous savons que les prochaines élections constitueront une étape décisive pour le destin de l'Union européenne du XXI siècle. groupe, engagé dans le projet européen, tient à réaffirmer à cette occasion l'urgence, répétée maintes fois dans cette enceinte, de renouer la confiance avec les peuples et d'en finir avec une technocratie qui discrédite et qui disqualifie l'idéal européen. Le Brexit, comme la montée des populismes, nous rappelle à nos responsabilités de politiques vis-à-vis des générations à venir. L'Union européenne doit être celle de la démocratie par et avec les peuples, disait le président Macron, sinon si elle prend le risque de ne plus être ! Très bien

Madame la présidente, madame la ministre, monsieur le rapporteur, mes chers collègues, notre commission spéciale a conduit un travail important, dans un délai très court, pour permettre au Sénat de se prononcer dans de bonnes conditions sur ce projet de loi d'habilitation.

aussi une aberration géostratégique, je le dis depuis deux ans. Après plus de quarante ans d'imbrication et de convergence, il nous faut travailler à la désimbrication et apprendre à gérer la divergence avec le moins de dégâts possible. Nous devons, par ailleurs, faire face à la forte incertitude qui pèse sur l'issue des négociations d'un accord de retrait. Nous avons reçu l'ambassadeur de Grande-Bretagne en poste à Paris. en avons conclu que la situation restait, à ce stade, encore très figée. La question irlandaise demeure le noeud gordien de la discussion. Le Sénat, au travers de son groupe de suivi commun aux commissions des affaires européennes et des affaires étrangères, que je copréside avec Christian Cambon, avait, à juste titre, tiré le signal d'alarme en juillet dernier. Il avait, en particulier, insisté sur la question irlandaise. Malheureusement, ses craintes d'un risque d'absence d'accord de retrait se révèlent, à ce jour, fondées. Je retiens également des propos de l'ambassadeur un message positif et rassurant sur la situation des Français

Nous devons donc nous préparer à toutes les hypothèses, y compris celle de l'absence d'un accord sur les modalités de retrait. C'est ce qu'entend faire le Gouvernement par le projet de loi d'habilitation qu'il a soumis au Sénat. Les mesures à prendre ne sont pas seulement d'ordre législatif beaucoup d'entre elles relèveront de l'Union européenne ou seront d'ordre réglementaire. Parallèlement, un travail préalable doit être conduit par les acteurs publics ou privés concernés. L'audition par la commission spéciale des représentants des activités portuaires, logistiques et de transport routier a bien montré les difficultés à surmonter.

Nous souhaitons que les administrations apportent tout leur soutien aux acteurs économiques qui vont faire face au Brexit. Il s'agit, madame la ministre, d'un enjeu de compétitivité pour notre pays, tout particulièrement pour nos ports, qui doivent relever un défi majeur.

Les grandes institutions du secteur des deux côtés de la Manche sont liées par quarante ans de régulations complexes. Dans ses deux rapports, le groupe de suivi avait signalé que, en quittant l'Union européenne, le Royaume-Uni devrait renoncer au passeport financier, qui permet à ses entreprises de vendre de vendre leurs services dans ce domaine dans le reste de l'Europe. D'autres questions juridiques se posent. Souvenons-nous que l'incertitude peut créer des risques majeurs pour les marchés financiers. Pour ce qui est du volet législatif, notre commission spéciale a veillé à ce que l'habilitation que le Gouvernement sollicite du Parlement soit précise. C'est une exigence constitutionnelle. Nous avons également fait attention à conforter les droits des personnes concernées par le Brexit. Ce faisant, nous n'avons pas écarté le besoin de flexibilité, imposé par l'incertitude même qui plane sur l'issue des discussions avec le Royaume-Uni. Le contenu des ordonnances sera, par ailleurs, subordonné

la France devra, en effet, rechercher une harmonisation avec les grands États membres voisins, en particulier avec l'Allemagne. Le rapport écrit expose les mesures prises par nos partenaires européens. Bien évidemment, le Sénat restera très vigilant quant à la suite du processus. C'est pourquoi nous avons souhaité que le Parlement puisse être saisi rapidement des projets de loi de ratification, pour se prononcer sur le contenu des ordonnances. Le groupe de suivi, que je copréside avec Christian Cambon, poursuivra ses travaux. Comme il l'a fait au cours des derniers mois, il rendra compte au Sénat des nouveaux développements concernant le retrait du Royaume-Uni. Il s'attachera aussi à évaluer les impacts du Brexit sur nos concitoyens installés dans ce pays et sur les secteurs économiques intéressés. Madame la ministre, je voudrais conclure en insistant sur l'attitude

Le groupe de suivi du Brexit, que le président Larcher nous avait demandé de constituer dès juillet 2016, gardera la même position.

Les partisans d'une Europe à tendance fédéraliste piétinent la souveraineté des États membres pour imposer une sorte de pensée unique. Ainsi, le résultat de plusieurs référendums a été contourné par les tenants d'une telle conception, qui n'hésitent pas à bafouer la volonté des électeurs dès qu'elle ne va pas dans leur sens. République, M. Macron, est à la pointe de la coalition qui essaye de torpiller le Brexit en pourrissant la négociation. Il s'agit encore de désavouer le suffrage universel, en poussant les Britanniques à organiser un nouveau référendum. À la veille des élections européennes, le but est de faire croire à nos concitoyens que l'évolution vers une Europe fédérale serait l'unique solution possible pour l'avenir. Au lieu de saboter le Brexit, la France devrait plutôt réclamer sa juste part dans la répartition des sièges au sein du Parlement européen. Actuellement, chacun des 6 députés maltais représente seulement 69 352 habitants, alors que chacun des 74 députés français représente 883 756 habitants. Pis encore, en totale violation du traité de Lisbonne, le ratio d'habitants par siège de la France est nettement plus défavorable que celui de l'Allemagne. De plus, si les opposants au Brexit parvenaient à leurs fins, cette injustice au détriment de la France subsisterait. En effet, lors du Conseil européen du 19 juin 2018, le Gouvernement français a accepté qu'en cas d'abandon du Brexit, la répartition actuelle des sièges soit maintenue à notre détriment, bien qu'elle viole le traité de Lisbonne. Avant de prendre des ordonnances, il convient donc de défendre notre représentativité en exigeant le respect de ce traité.

de son annulation. Il prévoit en effet que, dans le cas où le Royaume-Uni ferait toujours partie de l'Union au début de la législature 2019-2024, le nombre de représentants au Parlement européen par État membre

peu probable. En tout état de cause, si le Royaume-Uni venait à demander l'annulation de son départ avant les élections européennes, la décision de 2013 deviendrait caduque

Sur le premier point, si nous comprenons la nécessité d'acter le retrait du Royaume-Uni, il serait inacceptable que les ressortissants britanniques sur notre territoire puissent pâtir des négociations en cours, alors que, dans le même temps, de nombreuses mesures fiscales sont adoptées dans notre pays afin de « renforcer l'attractivité financière de la place de Paris. » J'ai à l'esprit, en particulier, l'annonce de la suppression de la dernière tranche de la taxe sur les salaires afin d'attirer chez nous les de la City.

La parole est à Mme Fabienne Keller, Nous sommes amenés à examiner les dispositions en cas de. Le texte national est complémentaire d'un texte européen, qui lui-même n'est pas encore connu. Mes chers collègues, comment en sommes-nous arrivés là ? Le choix des Britanniques du 23 juin 2016 nous conduit à réfléchir sur ce qui s'est passé. Je rappelle que ce vote a fait suite à plusieurs années de débats approfondis parmi le peuple britannique sur la question européenne. J'en tirerai deux leçons. Premièrement, la difficulté de l'Union européenne à prendre suffisamment en compte la demande des populations, l'appel, le besoin de liberté, le désir de souplesse face à ce qui est trop souvent perçu comme le carcan technocratique de Bruxelles.

L'Europe doit être demain plus déterminée que jamais sur les sujets à propos desquels elle est puissante, tout simplement parce qu'on est plus forts ensemble : je pense aux questions migratoires, mais aussi aux questions de défense ou encore aux questions de lutte contre le terrorisme. L'Europe demain,

Nous voilà, mes chers collègues, amenés à préparer l'hypothèse d'un, que nous souhaitons tous ne pas voir appliqué. Je salue le travail de la commission spéciale, de son président, de son rapporteur sur la question des droits sociaux et professionnels. Cette commission nous a aussi permis de mesurer les enjeux pour les ports, le commerce, l'économie, mais rien n'est joué. Nous espérons que ce texte ne sera pas appliqué. Nous n'oublions pas que les Britanniques sont de grands alliés et de grands partenaires. Je pense à la dernière guerre mondiale. Nous partageons aussi la volonté britannique de maintenir la paix en Irlande du Nord, c'est la dernière paix en Europe. Enfin, nous approuvons le souhait maintes fois exprimé de Michel Barnier

et droit à la libre circulation pour celles et ceux qui viennent passer quelques moments dans notre pays. Au regard de notre histoire commune,

mais aussi ceux qui décideront de revenir -puissent bénéficier des mêmes garanties. La deuxième question que je souhaitais évoquer concerne le sujet fondamental des activités économiques.

dont 2,5 milliards d'euros au titre des produits agroalimentaires et agricoles. Le Royaume-Uni est notre troisième client en matière de produits agroalimentaires et notre deuxième fournisseur de produits halieutiques,

ici même de démocratie. J'ai un tout autre regard sur ce référendum. On dit que les Britanniques ont voté pour la sortie de l'Union européenne, mais de quels Britanniques s'agit-il ? Je vous rappelle que des Jamaïcains, des Pakistanais, des Néozélandais, des Australiens ont pu voter

ce vote, pour beaucoup d'entre nous, constitue un déni de démocratie. Un tel sujet a été discuté pendant une campagne de six semaines

Deux conceptions de l'Europe s'opposent : d'une part, une Europe des nations respectant la souveraineté des états membres et les choix de chaque gouvernement démocratiquement élu d'autre part, une Europe à tendance fédéraliste qui piétine la souveraineté des états membres pour imposer la pensée unique des pseudo-élites. Le résultat de plusieurs référendums a déjà été contourné par les tenants de cette pensée unique, qui n'hésitent pas à bafouer la volonté des électeurs dès qu'elle ne va pas dans leur sens. Aujourd'hui, le Président Macron est à la pointe de la coalition qui essaye de saboter le Brexit en pourrissant la négociation. Là aussi, il s'agit de désavouer le suffrage universel en poussant les Anglais à organiser un nouveau référendum. À la veille des élections européennes, le but est de faire croire à nos concitoyens que l'évolution vers une Europe fédérale serait la seule solution possible pour l'avenir. MM. Macron, Juncker et Barnier sont-ils de bonne foi lorsqu'ils prétendent négocier des conditions loyales et honnêtes de sortie, alors que dans le même temps ils exigent la création d'une frontière douanière à l'intérieur du Royaume-Uni pour en disjoindre l'Irlande du Nord ? machiavélique que si demain l'Europe demandait à la France de créer une frontière douanière à l'intérieur de notre territoire, par exemple en séparant l'Alsace-Lorraine. Tous les problèmes qui justifieraient des mesures prises en urgence par ordonnance sont manifestement dus à la mauvaise volonté des responsables de l'Union européenne et à l'action du Président Macron, qui a organisé une véritable une véritable coalition pour essayer de pourrir les négociations sur le Brexit. On ne doit pas cautionner cette politique où quelques tenants de la pensée unique se targuent de donner des leçons de démocratie à des pays tels que la Hongrie ou l'Italie, dont les gouvernements sont pourtant élus de manière parfaitement démocratique.

celui de quitter l'Union européenne. Le sénateur Olivier Cadic le regrette, mais c'est un choix que nous respectons. Notre objectif est de mettre en oeuvre ce retrait ordonné du Royaume-Uni en préservant nos intérêts. Vous avez parlé de l'Irlande. l'Irlande. La position commune entre le négociateur britannique et l'Union européenne, que l'on retrouve dans le rapport conjoint de décembre 2017, 2017, consiste à éviter la mise en place d'une frontière physique entre les deux parties de l'Irlande. C'est un engagement qui a été confirmé par Mme May, dans une lettre adressée à Donald Tusk le 19 mars 2018. Cet engagement doit maintenant se traduire concrètement par une solution opérationnelle, juridiquement solide, dans le protocole à l'accord de retrait relatif à l'Irlande du Nord. Rien de plus, rien de moins Comme l'a signalé à plusieurs reprises Michel Barnier, il ne s'agit aucunement d'instaurer une frontière entre l'Irlande du Nord et le reste du Royaume-Uni, mais il s'agit de permettre les vérifications nécessaires pour préserver l'intégrité du marché unique et de l'union douanière, et par conséquent nos intérêts. nos intérêts. Un travail a été mené pour rendre les contrôles les moins contraignants possible. Je rappelle qu'il existe déjà des contrôles entre l'Irlande du Nord et le reste du Royaume-Uni.

qu'en dernier ressort et si aucune autre solution n'est trouvée dans le cadre de la relation future. C'est tout l'enjeu de la négociation qui a lieu actuellement, et c'est également toute la difficulté. Mais nous devons protéger

Mme la ministre. Cet amendement vise à ne pas couvrir dans le champ des mesures qui seront adoptées les ressortissants britanniques qui arriveraient en France après le le retrait britannique et à supprimer la reconnaissance immédiate des qualifications professionnelles des ressortissants britanniques qui exerceraient une activité en France au 30 mars. La commission spéciale souhaite que le texte cible également les salariés appelés à exercer leur activité en France au sein d'entreprises britanniques ayant fait le choix de s'y déployer après le retrait du Royaume-Uni, afin notamment de renforcer l'attractivité de la France. L'amendement proposé vise à ne pas couvrir ces salariés.

». Les Britanniques qui arriveront après le 31 décembre 2020 ne sont actuellement pas couverts par l'accord de retrait tel qu'il est négocié. L'article 9 du projet d'accord de retrait, qui est agréé entre les négociateurs, stipule en effet que seuls sont couverts par l'accord de retrait les ressortissants britanniques qui vivent dans un État membre avant le 31 décembre 2020. Dans ces conditions, la rédaction actuelle du texte équivaudrait à prévoir un régime plus favorable pour les ressortissants britanniques en l'absence d'accord de retrait qu'en cas d'accord de retrait.

prévoir pour les ressortissants britanniques un statut plus favorable que celui qu'il a su négocier dans le projet d'accord de retrait, qui est aujourd'hui presque finalisé. Le faire, ce serait encourager

La commission spéciale souhaite préciser la finalité de la clause balai, prévue à l'article 1, en précisant qu'elle vise à « préserver les intérêts de la France en matière économique, financière, de défense et de sécurité Une telle rédaction réduit significativement le champ des mesures qui pourraient être adoptées, et donc l'utilité de cette clause balai dont la rédaction telle qu'elle était proposée par le Gouvernement avait été validée par le Conseil d'État. L'amendement n° 12 vise donc à prévoir une finalité suffisamment large pour permettre l'adoption de l'ensemble des mesures nécessaires à l'égard des ressortissants britanniques, un de nos objectifs étant, par exemple, la préservation des intérêts des ressortissants français au Royaume-Uni.

Le Gouvernement a l'obligation d'indiquer avec précision au Parlement quelle est la finalité des mesures qu'il se propose de prendre et leur domaine d'intervention Dans son avis, le Conseil d'État, lui, a appelé le Parlement à jouer son rôle et à préciser l'habilitation tout en laissant suffisamment de flexibilité au Gouvernement.

Mme la ministre. Cet amendement vise à préserver une finalité suffisamment large pour tenir compte, lors de l'adoption des mesures, de l'issue des négociations et de l'adoption par le Royaume-Uni de mesures réciproques. La commission spéciale a souhaité préciser la finalité des ordonnances prévues à l'article 1. Cette rédaction n'est cependant pas satisfaisante, car elle ne préserve pas la possibilité pour le Gouvernement de tenir compte de l'adoption de mesures équivalentes de l'adoption de mesures équivalentes par le Royaume-Uni à l'égard des ressortissants français ou de mesures prises par les autres États membres. Une rédaction alternative est en conséquence proposée de façon à marquer une direction

ce qui- ne nous mentons pas -sera sans doute hors d'atteinte. Il y aura des conséquences au Brexit. Dire que l'on est capable de préserver totalement ou de garantir absolument les activités économiques ou le sort des ressortissants britanniques sur notre territoire est une illusion.

imprécisions ou accusations sans y répondre. Nous avons souhaité ne pas mentionner seulement les contrôles sanitaires et phytosanitaires, d'une part, parce qu'ils sont déjà mentionnés

des consommateurs et du secteur agricole. C'est le premier sujet dont je me suis entretenu avec le nouveau ministre de l'agriculture lorsqu'il a pris ses fonctions. Je lui ai demandé s'il considérait que les effectifs prévus étaient suffisants.

par l'ensemble des ministères et des administrations. Et pourtant, c'est une réalité ! Mais telle est la vie du dialogue entre le Gouvernement et le Parlement ... J'approuve, dans la nouvelle rédaction, la mention des accords bilatéraux, la référence aux accords de retrait

demeure problématique selon le Gouvernement. En effet, les ordonnances pourront prévoir des mesures temporaires, mais non pas régler la situation en France des ressortissants britanniques. Là encore, prétendre que l'on va préserver

dans le cadre des négociations que l'Union européenne et vous-même menez avec nos amis britanniques, et celle qui est retenue par M. le rapporteur, qui vise à répondre au mieux aux préoccupations exprimées par le Conseil d'État,

à Mme la ministre. Cet amendement vise à préciser le type de modalités envisagées pour les ordonnances, tout en permettant l'adoption de l'ensemble des mesures nécessaires. La commission spéciale a souhaité préciser la finalité des ordonnances prévues à l'article 1, qui doivent viser « à prévoir des dérogations, des procédures administratives simplifiées et des délais de régularisation pour les personnes morales ou physiques concernées ». Une telle rédaction ne permettrait pas de couvrir l'ensemble des mesures envisagées, et notamment pas la mise en place d'un régime juridique allant au-delà des simples dérogations. La rédaction proposée vise en conséquence à couvrir des dérogations, mais également les adaptations de la législation de droit commun, ce qui peut inclure des régimes spécifiques, et nous n'avons pas de raison de l'exclure aujourd'hui. Quel est l'avis de la la commission spéciale ? Une fois de plus, la commission est plus précise que le Gouvernement. Vous évoquez, madame la ministre, la possibilité de créer des procédures administratives pour

L'alinéa 16 prévoit la possibilité pour le Gouvernement de suspendre l'application des mesures prévues par les ordonnances prises en application du présent article s'il venait à constater que le Royaume-Uni n'accorde pas un traitement équivalent aux ressortissants français au Royaume-Uni. Une telle suspension devra prendre effet à compter d'une date prévue par décret, qui sera expressément précisée dans les ordonnances. Néanmoins, dès lors qu'il s'agira pour le Gouvernement de suspendre par décret des mesures qui sont de nature législative, une telle habilitation doit expressément être prévue par le législateur, et donc figurer dans la loi d'habilitation. C'est ce que nous vous demandons de voter, car elle ne peut être prévue seulement au stade de l'ordonnance.

à habiliter le Gouvernement à légiférer par ordonnances. L'habilitation ne renvoyait à aucun décret. Pourtant, dans l'ordonnance du 22 septembre 2017, le Gouvernement a renvoyé à des décrets pour fixer les conditions d'application des mesures, en particulier aux articles 4, 8, 10, 16, 20, 24, 28, 33, 37, 38 et 40. Je croyais que

Si aujourd'hui la plus grande incertitude subsiste au sujet des modalités du Brexit, c'est parce que, au sein de l'Union européenne, beaucoup de responsables font tout leur possible pour compliquer les négociations. En fait, ils souhaitent punir les Britanniques d'avoir décidé de sortir de l'Union européenne. Ils pensent en effet que plus les Britanniques rencontreront de difficultés, plus nos concitoyens accepteront l'idée que l'évolution vers une Europe fédérale serait la seule solution pertinente pour l'avenir. Manifestement, ils ne sont pas de bonne foi lorsqu'ils prétendent négocier des conditions loyales et honnêtes de sortie, alors que dans le même temps ils exigent la création d'une frontière douanière à l'intérieur du Royaume-Uni pour en disjoindre l'Irlande du Nord. Ce projet de loi sur les ordonnances n'est théoriquement justifié que par l'urgence. C'est donc la conséquence directe du retard pris par les négociations du Brexit, lequel résulte lui-même des exigences volontairement extravagantes formulées par l'Union européenne.

des ressortissants français au Royaume-Uni, des autorités britanniques. L'objectif de cet alinéa est de permettre la portabilité des droits sociaux et la prolongation des droits professionnels, dont la liste a déjà été dressée au I Il est cependant malaisé de l'écrire juridiquement de façon concise, sans risquer de couvrir un champ insuffisamment large. C'est la raison pour laquelle le Gouvernement propose de faire une référence explicite aux situations « dans les champs visés aux 1° et 2° du I ».

concerne les ports, la majeure partie des échanges entre le Royaume-Uni et le continent passe par le nord de la France. Les chiffres pour 2017 du trafic franco-britannique dans la zone de Calais et de Dunkerque parlent d'eux-mêmes : plus de 30 millions de passagers, 4,2 millions de poids lourds, 73 000 autocars traversent la Manche par les ferries, et 51 000 autocars empruntent le tunnel. ce sont 745 millions de tonnes de marchandises qui ont transité par les ports du nord de la France. À cela s'ajoute le fret express- je pense à Amazon ou à eBay -, qui passe par le Royaume-Uni avant d'arriver sur le continent. Or, aujourd'hui, les ports français n'ont ni la place ni les équipements pour effectuer les contrôles douaniers de poids lourds. Encore une fois, si nous comprenons la nécessité d'assouplir le droit existant afin de de répondre à l'urgence, il faut noter que les moyens financiers manquent. Cela n'est pas nouveau : la Cour des comptes, faisant dans son rapport annuel de 2017 le bilan de la réforme portuaire de 2008, pointait, en dehors de la question du Brexit, la faiblesse de nos ports, liée à un manque de vision claire mais surtout d'investissement. Elle rappelait que la répartition des crédits de l'État devrait cibler les investissements dans les grands ports maritimes soumis à un réel enjeu de compétitivité à l'égard des ports voisins de la mer du Nord. Bien qu'il s'agisse d'un enjeu national important, cela n'a pas été fait. C'est cette inaction de l'État que nos ports paient aujourd'hui. Dès lors, comment expliquer que le Gouvernement n'ait pas jugé nécessaire de prévoir un fonds de réserve spécifique pour parer au défi logistique du Brexit, à l'image de ce qui a pu être fait au Danemark, par exemple ? L'amendement

Mme la ministre. Cet amendement vise à rétablir la mention du « notamment », précédemment évoquée par le rapporteur, avant la liste des domaines qui pouvaient être concernés par des adaptations ou des dérogations. Une telle mention est indispensable pour permettre l'adoption de l'ensemble des mesures qui pourraient être nécessaires, tout simplement parce que nous sommes dans un exercice totalement inédit. les enjeux soulevés par le retrait britannique avec beaucoup de volontarisme depuis des mois puisque, depuis le mois d'avril, le Premier ministre a demandé à l'ensemble des administrations de travailler sur les conséquences d'un éventuel dans le dans le cas du Brexit. Il n'est pas possible, à l'heure actuelle, de réaliser un travail totalement exhaustif de recensement des adaptations qui pourraient être nécessaires. nécessaires. La modestie nous oblige à le dire, il serait arrogant de notre part de prétendre que nous savons absolument tout dans le détail. C'est notamment le cas pour les aménagements dans les ports, lesquels étaient habitués à gérer du commerce intracommunautaire et sont aujourd'hui confrontés à des problématiques nouvelles. J'ajouterai que nous devons veiller à rester compétitifs face aux adaptations qui seront prévues par les autres États membres concernant « notamment » leurs installations portuaires.

Je vous rappelle, mes chers collègues, que l'article 3 permet d'adapter le droit en vigueur concernant l'aménagement,

s'adapteront sans difficulté : leurs trafics sont internationaux et les quelques aménagements qu'ils devront réaliser se feront vraisemblablement sans qu'il y ait de problème au regard de leur capacité financière, de leur disponibilité foncière et de leur expertise technique. Je suis beaucoup plus inquiet pour les ports de plus petite taille. Je prendrai l'exemple que je connais le mieux, celui de Dieppe en Seine-Maritime,

les premières estimations d'investissements à réaliser pour améliorer les capacités de stockage, permettre les aménagements nécessaires à l'arrivée d'agents des douanes, exercer les contrôles phytosanitaires s'élèvent à plus de 3 millions d'euros.

les difficultés qui pourraient être engendrées par les délais de l'autre côté et par la question, qui n'a pas été évoquée ici mais qu'il faudra bien traiter, des migrations, des migrations irrégulières qui empruntent ces flux de transports, la situation risque d'être extrêmement difficile. Ce texte est donc important. Il faudra que le Gouvernement,

du port de Dunkerque, du port du Havre et de Ports normands associés, c'est-à-dire Cherbourg, Caen et bientôt Dieppe. Effectivement, la partie sera rude pour certains de ces ports.

de loi présenté par le Gouvernement prévoyait un délai de six mois, qui a déjà été ramené à trois mois sur proposition du rapporteur de la commission spéciale. Or le Gouvernement fait preuve d'une évidente désinvolture à l'égard du Sénat, que ce soit en refusant de lui communiquer l'avis du Conseil d'État sur le projet de loi initial ou en proposant des articles délibérément flous et imprécis, ce que le Conseil d'État a d'ailleurs déploré.

quel que soit le délai. Je veux rappeler des chiffres qui figurent dans mon rapport : pour la session 2016-2017, des projets de loi ont été déposés au Sénat pour ratifier 71 ordonnances.

six mois, plus long que le délai habituel de trois, pour une véritable raison. Ce délai est en effet nécessaire pour permettre au Gouvernement de présenter au Parlement, qui y tient et je le comprends, un projet de loi qui tirera les conséquences des premiers mois de mise en oeuvre des ordonnances, notamment- ce point a été mentionné la mise en oeuvre par le Royaume-Uni de mesures réciproques. L'une des spécificités de notre approche est que le Gouvernement s'assurera de la réciprocité des mesures prises par le Royaume-Uni. L'alternative reviendrait à présenter un projet de loi de ratification qui aurait de très grandes chances de devoir être modifié à brève échéance par le Gouvernement. C'est la raison pour laquelle je donne un avis défavorable à cet amendement. Vous l'aurez sans doute deviné, mesdames, messieurs

extrêmement réactifs, attentifs et aux côtés des entreprises françaises. Mes chers